Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui a pour vocation d'éclairer le rôle que doit jouer l'État dans la définition de notre politique industrielle. Cette question, centrale en temps normal, devient essentielle en temps de crise. Depuis un an, l'épidémie de covid-19 agit comme un révélateur des failles de notre société ; les fragilités de notre modèle industriel sont apparues en pleine lumière quand il a fallu faire face à des pénuries de produits qui, seuls, pouvaient nous permettre de lutter contre la maladie. L'épreuve que nous traversons a néanmoins un intérêt : elle remet enfin au centre du débat public la question de la reconquête industrielle. C'est donc notre conception de la souveraineté nationale dans ce domaine qui est interrogée.

Le 30 août dernier, Veolia, numéro un français de la gestion de l'eau et des déchets, annonce son intention de racheter le numéro deux, Suez, son concurrent historique, en se portant candidat à l'acquisition des parts qu'Engie avait annoncé céder.

Depuis le départ, je vous le dis franchement, monsieur le ministre, la position de l'État n'est pas claire. La rapidité de l'offensive menée par Veolia interroge. Vous me répondrez que vous avez oeuvré pour qu'un délai supplémentaire soit accordé afin que Suez puisse soumettre une offre alternative. Certes.

tant les autres parties, qui auraient pu rejoindre leur position, ont fait basculer très opportunément le vote final en s'abstenant ou en quittant la salle. Pouvons-nous, pouvez-vous, accepter un tel camouflet ? Aujourd'hui, Veolia détient 29,9 % des parts de Suez. Encore récemment, la proposition des dirigeants de Suez en date du 21 mars dernier a été rejetée par Veolia et la voix de l'État n'a pas été entendue, alors que cela aurait pu aboutir au rapprochement amical que vous appelez de vos voeux.

Si vous ne représentiez qu'un actionnaire privé, monsieur le ministre, les marchés vous auraient sanctionné après avoir constaté la faible efficacité de votre action et le manque de rentabilité de votre travail. Or vous n'êtes pas un actionnaire comme les autres : vous représentez l'intérêt général.

À ce stade, nous constatons que ces conditions ne sont pas remplies. À ce stade, vous n'avez pas été en mesure d'apporter des garanties à la représentation nationale, pas plus- c'est peut-être plus grave -qu'aux salariés concernés. Comment pouvez-vous nous garantir que cette OPA n'emportera pas de conséquences sociales, environnementales et territoriales qui affecteraient durablement notre pays ?

Comment pouvez-vous nous garantir que la compétitivité d'un nouveau groupe d'une telle taille ne soit pas fortement menacée ? Comment pouvez-vous nous garantir que cela ne favorisera pas l'apparition d'acteurs défendant un moins-disant social ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'OPA se voulait amicale, mais les hostilités ne cessent pas, dans un contexte pandémique provoquant des incertitudes financières. Était-il vraiment opportun pour le groupe Engie de vendre ses participations dans Suez ? Le Gouvernement a, semble-t-il, désapprouvé ce mouvement dans un premier temps, alors que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a salué, par la voix de son directeur général, une « OPA amicale », rompant ainsi avec sa neutralité classique. Faut-il le rappeler ? La CDC pèse 10 % des droits de vote au sein de Veolia. Pourtant, son conseil de surveillance n'a pas donné son avis sur cette opération. Toujours est-il que les 18 euros de l'offre d'achat initiale sont désormais le niveau atteint par l'action de Suez, ce qui laisse rêveur quant aux dernières spéculations.

Collectivités locales et territoriales, syndicats, régies font maintenant face à l'incertitude sur les évolutions et les dévolutions du marché. La séquence pose question pour de nombreux décideurs. Elle crée, sans aucun doute, un appel d'air sans précédent pour les concurrents intermédiaires, soucieux de peser davantage et dans l'attente de cessions d'actifs imposées par les autorités.

À l'inverse, la séquence renforcera la financiarisation des deux opérateurs, alors qu'il faudrait un ancrage actionnarial portant une vision à long terme. Le risque de l'entrée de fonds activistes et purement spéculatifs est réel et inquiétant. Engie aurait pu développer des coopérations industrielles mariant des compétences énergétiques et environnementales en travaillant sur la numérisation des données dans une approche de très attendue. Le groupe a préféré vendre, une stratégie peut être plus politique qu'industrielle. Quelles seront les incidences de ces évolutions sur l'ensemble des usagers, sur les collectivités locales et territoriales et sur les syndicats ? Prenons un exemple en tenant compte des concentrations actuelles. En remportant la délégation du service public pour la gestion de l'ensemble des incinérateurs de la métropole bordelaise, Veolia a implicitement créé un différentiel de prix important entre la métropole et le reste du département, dans un marché captif en raison de l'absence de concurrence. À l'heure des coopérations territoriales, c'est un exemple provocant. Suez multiplie aujourd'hui les projets de cessions ; Veolia y voit une volonté d'amplifier les dividendes pour consolider sa majorité et sa gouvernance dans la tempête actuelle, mais ni les usagers, ni les collectivités, ni les salariés n'en sortiront gagnants. Il faut siffler la mi-temps, mais comment finir le match ? Monsieur le ministre, le souhaitez-vous ? En avez-vous les moyens ? La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la position de l'État sur Veolia et Suez a été constante : nous souhaitons que cette opération se fasse dans un cadre amiable, nous refusons que le conflit l'emporte sur le dialogue et nous refusons la guerre de tous contre tous, qui ne fera que des perdants. Pour répondre à la question de Patrick Kanner, pour décider de soutenir ou non la cession par Engie de sa participation dans Suez à Veolia, puisque l'État est actionnaire- actionnaire minoritaire, la pérennité de l'emploi- sujet évidemment majeur -, la logique industrielle, la préservation d'une offre concurrentielle, essentielle pour les collectivités locales auxquelles vous êtes particulièrement attachés, l'intérêt l'intérêt patrimonial, l'État étant actionnaire d'Engie. Veolia a pris un certain nombre d'engagements sur ces points, notamment sur l'emploi, sur l'investissement et sur le maintien de la recherche et du développement en France. J'ai toutefois toujours été très clair sur le fait que sur le fait que cette opération devait être amicale, c'est-à-dire acceptée par le conseil d'administration de Suez et par l'ensemble des parties prenantes. Dans cette affaire, monsieur le sénateur, j'ai pris mes responsabilités. Dès lors que cette offre n'était pas acceptée par le conseil d'administration de Suez, j'ai demandé que le représentant de l'État au conseil d'administration (CA) d'Engie vote contre la cession des participations d'Engie dans Suez.

en dehors des entreprises plutôt que l'intérêt général dans les entreprises, sauf pour des services publics ou certaines entreprises stratégiques. C'est la position constante que je défends depuis quatre ans que je suis ministre de l'économie, des finances et de la relance et cette affaire n'a fait que me conforter dans cette conviction

garantir l'attractivité de notre territoire, pour faciliter le financement de l'innovation et de la recherche qui fera la puissance de la nation française et de l'Europe au XXI siècle. De ce point de vue, je tire quatre leçons de la crise actuelle pour la définition de la place de l'État dans l'économie.

Toutes les décisions que nous avons prises- baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse de l'impôt de production, indispensable pour l'attractivité industrielle du pays -, tous les choix que nous avons faits avec le Président de la République depuis 2017 nous ont permis

et elle est vitale au lendemain de cette crise où les innovations technologiques vont s'accélérer, est de financer les investissements dans l'innovation, de faire le choix des innovations de rupture, de soutenir sans cesse l'investissement, l'investissement et toujours plus d'investissement.

nous ont permis de définir un certain nombre de nouvelles filières dans lesquelles la France va investir : l'hydrogène, le calcul quantique, les biotechnologies, l'agroalimentaire,

et c'est pourquoi nous négocions pied à pied avec la Commission européenne une réforme d'EDF qui maintienne l'unité de cette grande entreprise énergéticienne. Je veux Je veux le dire à cette tribune avec beaucoup de force : nous refuserons tout démantèlement d'EDF. Nous voulons la transformer pour qu'elle investisse davantage, notamment dans les énergies renouvelables, et cela peut se faire en maintenant l'unité du groupe. Avec le Président de la République, c'est notre ambition. Enfin, la quatrième responsabilité de l'État, c'est de protéger : protéger nos technologies, nos savoir-faire, notre indépendance. Ne soyons pas naïfs sur le monde dans lequel nous entrons.

est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'idée que nous nous faisons de l'État dans l'économie. Il a un rôle essentiel à jouer, mais celui-ci doit être clairement défini : créer un environnement favorable à l'investissement, encourager l'innovation, préserver nos services publics, protéger nos technologies de pointe. Voilà ce à quoi je m'attache depuis près de quatre ans.

de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires,

en charge notamment du contrôle des autorités exécutives, de nombreuses questions demeurent sur l'attention et l'action des pouvoirs publics et de l'État actionnaire. Nous avons constitué ici

Ils sont présents, l'un et l'autre, dans des activités qui sont à maturité sur le marché français et, pour se développer et rester compétitifs, ils doivent bénéficier de la dynamique du marché mondial. Le risque est grand, pour l'entité dont les activités seraient principalement circonscrites à la France, de voir sa pérennité remise en cause Quel avenir, en cas de fusion, pour la part de ces activités jugées moins stratégiques et cédées ? Même si celles-ci échappaient à la vente à la découpe, quelle dynamique interne auront-elles, coupées des activités avec lesquelles elles développaient des synergies ? Depuis la fin de l'été 2020, l'annonce de la vente des parts d'Engie dans Suez a été suivie de déclarations parfois discordantes au sein de l'État. Quelle était alors réellement la stratégie de l'État actionnaire et de son levier opérationnel qu'est l'Agence des participations de l'État a-t-elle fait connaître à Engie des demandes particulières en termes de dividendes ou de valorisation boursière ? Comment l'État actionnaire entend-il agir désormais pour réussir sa médiation et assurer le développement, à l'international et en France, de groupes français performants, efficaces, offrant un service essentiel à à nos concitoyens

je ne veux pas et je ne peux pas croire un instant que, dans les dernières années, le sort de Veolia et de Suez, deux pépites françaises de surface mondiale, fussent-elles des entreprises privées,

pour ces deux groupes ? Pire, que l'État n'a pas su jouer son rôle et insister auprès de Veolia et, comme l'a dit Patrick Kanner, auprès d'Engie, pour permettre l'émergence d'offres alternatives La précipitation des acteurs et la contradiction apparente au sein même de l'État n'ont pas permis de prendre ce recul. Quelle destruction de valeur en seulement quelques semaines !

à son détriment et au détriment des collectivités territoriales. Votre politique étant de permettre l'investissement, l'investissement et l'investissement, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, vous devez jouer un rôle dans ces négociations.

à ses effets et accepter un bazar pareil entre deux entreprises majeures stratégiques de l'environnement. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Il existe encore une fenêtre d'opportunité jusqu'au 20 avril prochain, qui permet une médiation de l'État. Comment vos services sont-ils mobilisés pour faire aboutir une solution concertée, ambitieuse et pérenne ? Vous avez raison, l'important, c'est la vision que nous partageons sur ces services fondamentaux de l'environnement. La parole est à M. le ministre.

privées. Notre souhait était de permettre à Engie de se développer et de se recentrer sur ses activités ; chacun sait qu'elle gérait un portefeuille d'activités trop diversifié et qu'il lui était nécessaire de simplifier et de clarifier sa stratégie industrielle.

est oui. L'a-t-il fait ? Oui, nous l'avons fait au début et nous avons continué à le faire au cours des dernières semaines, puisque j'ai souhaité que le directeur général du Trésor lance

j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en appeler à la renaissance d'un véritable ministère de l'industrie, c'est-à-dire d'un ministère exclusivement chargé de concevoir et d'appliquer une stratégie industrielle pour notre pays. Je me réjouis que nos collègues socialistes, conscients de la nécessité de conserver le patrimoine industriel français, aient inscrit ce débat à l'ordre du jour. Malheureusement, auparavant beaucoup de gouvernements ont laissé des rachats de nos fleurons se faire, entraînant la perte progressive d'un précieux savoir-faire industriel.

Afin de préserver les emplois, et surtout de maintenir les compétences industrielles de notre pays, le Gouvernement s'emploie- il faut le saluer -à créer de nouvelles chaînes de valeur. Au-delà de son rôle dans le développement d'une stratégie de long terme, l'État doit être également attentif aux prises de contrôle des entreprises françaises et sauvegarder nos savoir-faire technologiques. Si l'OPA lancée par Veolia sur Suez aboutissait, elle aurait pour effet de fusionner l'activité internationale de deux champions français. Pourtant, certains exemples de fusion soulèvent la difficulté des restructurations qui les suivent. Au-delà de cette opération, plusieurs questions se posent. Estimez-vous, monsieur le ministre, qu'un rapprochement de ce type met par principe en péril le patrimoine industriel français ? Le Gouvernement a-t-il établi une liste des industries à valeur stratégique ? Quel est le plan d'action du Gouvernement pour les sauvegarder et les développer ? Quelle reconquête industrielle quelle articulation avec nos partenaires européens permettraient à nos entreprises de peser suffisamment sur la scène internationale, notamment des regroupements du type Airbus ? de la solidarité européenne quand nos partenaires polonais achètent des avions de chasse américains, ou quand nos partenaires allemands formulent des exigences au sujet du nouvel avion de chasse européen ? La parole ministre. Monsieur le sénateur, j'estime que peu de gouvernements se sont autant employés à protéger notre industrie

Nous sommes intervenus pour favoriser le rapprochement entre Alstom et Bombardier, qui permet de créer un leader dans le domaine de l'industrie ferroviaire. Je n'ai pas hésité- cela peut pourtant paraître surprenant de ma part -à nationaliser les Chantiers de l'Atlantique. Nous avons renoncé au rapprochement avec Fincantieri, de concert avec notre partenaire italien, parce que nous estimions que les conditions n'étaient plus remplies. Lorsque l'acteur canadien Couche-Tard- tout à fait respectable par ailleurs

un conflit ouvert entre deux géants industriels. Comme je l'ai indiqué clairement à la présidente Sophie Primas, nous sommes intervenus pour pacifier les choses et rapprocher les positions des deux parties. Je souhaite maintenant qu'elles écoutent

Cette bataille est devenue une véritable tragédie grecque à partir du moment où Engie a accepté l'offre d'achat proposée par Veolia malgré l'opposition de l'État actionnaire. D'un côté, Veolia veut créer en France le super champion mondial de la transformation écologique de l'autre, Suez, absolument opposé à tout projet de fusion dans les termes proposés par Veolia, s'alarme pour ses 90 000 collaborateurs, dont 30 000 en France, et évoque une menace de suppressions d'emplois. En sous-main, des fonds d'investissement gravitent autour des deux géants Meridiam, à proximité de Veolia, ne cesse de montrer patte blanche pour rassurer les salariés de Suez, tandis qu'Ardian et GIP, autour de Suez, affirment vouloir assurer l'indépendance et l'intégrité du groupe. entre ces deux géants, un grand nombre de communes françaises ne cachent pas leur inquiétude. Ce projet de fusion pourrait en effet concerner toutes les collectivités qui ont délégué la gestion de leur eau à l'un ou à l'autre de ces deux groupes. À ce jour, la situation paraît difficilement conciliable, et nous nous acheminons vers des enchères boursières. Pourtant, face à des enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux majeurs, notre État stratège doit conforter son rôle. Alors que la journée internationale de l'eau était célébrée le 22 mars dernier et qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, quelles autres possibilités s'offrent à nous pour régler une situation complexe, potentiellement préjudiciable en termes d'emploi, et dont l'issue doit apporter une réponse viable aux deux protagonistes et permettre à la France de gagner davantage de visibilité face à des concurrents étrangers toujours plus redoutables ? La parole

transformation des entreprises, ou loi Pacte. Après le rejet de cette réforme par le Sénat en 2018, un projet de référendum d'initiative partagée avait été proposé pour la première fois par des parlementaires, recueillant un peu plus d'un million de signataires. L'ironie de l'histoire veut que ce soit la crise du covid qui ait enterré ce projet contesté. Après une année de pandémie, ces débats paraissent anciens. Plus récemment, monsieur le ministre, vous avez pris la décision d'empêcher un projet de fusion entre l'entreprise Carrefour et le groupe de supérettes canadiennes Couche-Tard.

Le cas de Veolia-Suez est un peu différent, puisqu'il s'agit d'une offre publique d'achat entre deux entreprises concurrentes, mais françaises, dans un secteur qui intéresse de nombreux acteurs : entreprises, salariés, consommateurs et élus locaux. L'examen du projet de loi Pacte avait aussi été l'occasion de débattre de la notion d'entreprise stratégique et de renforcer les pouvoirs de contrôle du ministère de l'économie sur les autorisations d'investissements étrangers dans certains secteurs d'activité.

notre manière de vivre, la qualité de notre alimentation, notre sécurité sanitaire, et c'est bien ce qui est en jeu dans la grande distribution. En effet, les grands distributeurs français ont créé un modèle- ils peuvent en être fiers -d'approvisionnement auprès des filières agricoles françaises. Qui ici peut me garantir que le rachat de Carrefour

J'en félicite la direction et les salariés de Carrefour, car c'est bien la preuve que ce groupe a su se réinventer et innover au cours des derniers mois.

L'enjeu de la partie consiste à gérer la majeure partie de l'or bleu de notre pays, les déchets et les services à l'environnement indispensables pour assurer la transition écologique. Comment expliquer, comment croire que le projet d'absorption de Suez ait pu surprendre par sa rapidité d'exécution l'État, à la fois comme puissance publique et comme actionnaire d'Engie, mais aussi de Veolia, puisque la Caisse des dépôts et consignation en est le premier actionnaire ? Après Alstom, Nokia, Technip, Engie, General Electric, les Chantiers de l'Atlantique, la volonté de privatiser ADP et de casser EDF, nous assistons aujourd'hui au démantèlement d'un champion français

En revanche, cela ne vous dérange absolument pas que des monopoles privés se constituent au seul profit des actionnaires et au détriment des usagers, des salariés et des collectivités. Dès lors, la seule question est quand l'exécutif décidera-t-il d'arrêter la grande braderie afin de permettre à l'État de jouer son rôle de garant de l'intérêt général, de stratège et d'actionnaire ? En tant que bien commun,

Nous nous battons pour maintenir l'unité d'EDF, ce grand service public de l'énergie : vous devriez nous en être reconnaissants ! Non ! Nous nous battons aussi pour préserver le nucléaire. Je crois

nous sommes attachés à la constitution de champions nationaux et européens afin de peser sur la compétition internationale. est d'ailleurs le principal argument utilisé par les promoteurs de la fusion entre les entreprises numéro un et deux du secteur du retraitement des déchets et de l'eau.

leur droit de veto contre la fusion d'Alstom et de Siemens en février 2019. Il est rare que de tels mariages entre deux acteurs déjà champions dans leur domaine soient autorisés. Or trois arguments allant dans ce sens pourraient être pris en compte. Premièrement,

-, les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales, soulignent à raison les bienfaits de la concurrence en termes de prix et de qualité de service.

Alors que l'idée défendue par la France d'une réforme du règlement européen sur les concentrations n'est pas à l'ordre du jour, et alors que la méfiance européenne envers les grands groupes est bien d'actualité comme le démontre le cas d'EDF,

Il est donc légitime que je sois en contact régulier avec la Commission européenne sur ce point. Vous avez unanimement appelé à juste titre au maintien d'une saine concurrence dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau.

Depuis sept mois maintenant, les collectivités qui doivent renouveler leur contrat s'interrogent. Depuis sept mois maintenant, l'image des deux champions français s'abîme sur la scène internationale. Depuis sept mois, finalement, seuls les banquiers d'affaires et les avocats se frottent les mains. Il faut désormais sortir de cette crise collectivement. C'est pourquoi, cet après-midi, je vous propose modestement une solution de sortie de crise : demandons aux salariés de Suez, leur intersyndicale, de construire et de soumettre publiquement un cahier des charges aux actionnaires actuels et futurs. Ce cahier des charges porterait notamment sur les garanties sociales et sur les effectifs ; sur la participation des salariés au capital de l'entreprise ; sur l'investissement dans les activités et dans les métiers de demain la présence d'actifs en France et à l'international permettant d'assurer la pérennité et le développement du futur groupe Suez ; sur les activités sur tout le territoire, le partenariat avec les collectivités et le service aux usagers ; et enfin, sur la création d'une fiducie garantissant la tenue des engagements.

Gaulliste « canal historique »- vous me connaissez, monsieur le ministre -, je suis attaché au principe de l'intervention de la puissance publique quand il s'agit de défendre l'intérêt de la Nation et ce qui reste de son patrimoine industriel. Nous avons là deux champions européens dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets. Le respect de la juste concurrence permet aux collectivités de pouvoir les mettre en compétition pour leur délégation de services publics. Aujourd'hui, Veolia lance une OPA hostile sur le groupe Suez après avoir racheté 29 % du capital de cette société à Engie, avec la bénédiction du Gouvernement- ne vous en déplaise, nous expliquent que ce rachat déboucherait sur la création d'un « champion mondial » dans le domaine. Ne serait-il pas plus pertinent de garder deux champions nationaux, voire européens, comme le propose Suez, dans une solution qui serait négociée ?

À cette logique de fusion-absorption systématique, je préfère la saine concurrence qui renforce la créativité, l'innovation, et l'investissement massif en recherche et développement. Je ne prendrai que deux exemples. Comment contester le statut de leader des groupes LVMH et Kering, ou bien encore celui des groupes EDF et Engie, pourtant concurrents en France ?

Comment expliquer aux Français que l'État n'intervienne pas dans la cession des parts qu'Engie possédait dans Suez, ouvrant ainsi la porte à la fusion des deux sociétés, et que le Gouvernement réclame ensuite le maintien des deux leaders, la protection de l'emploi et la préservation intégrale de la concurrence ? toujours le « en même temps » ! Où est l'État stratège ? Monsieur le ministre, une bonne fois pour toutes, quelle est votre position sur ce dossier ? De gaulliste à gaulliste, monsieur Cadec, nous défendons la même position, celle de la préservation d'une concurrence entre deux champions industriels français. Comme je le dis depuis le début de ce débat, je pense que c'est la bonne option.

Une entreprise géante en situation de monopole aurait un pouvoir de marché très fort, trop fort pour de nombreuses collectivités délégataires dont elle serait le seul cocontractant possible.

Veolia a récemment proposé de céder les activités françaises de Suez en cas de fusion. Suez a commencé par faire état d'offres d'acquisition de ses activités françaises dans le domaine de l'eau et des déchets, de déclarer il y a quelques jours avoir rendu incessibles, par le biais d'une fondation, ses deux principales sociétés d'eau en France jusqu'en 2024. Veolia a alors saisi la justice. Au milieu de cette bataille juridique, financière et boursière, l'État paraît adopter une position de simple observateur et de nombreuses collectivités délégataires

Je rappelle également qu'au-delà de la médiation dont j'ai parlé à la présidente Sophie Primas, nous avons engagé un dialogue avec la Commission européenne, qui est chargée de l'examen de cette opération, au titre du droit de la concurrence. Je redis

Aussi, pour éviter cet écueil aux yeux des autorités de la concurrence, le rapprochement des deux entreprises permettrait de créer une nouvelle entité rassemblant l'ensemble des activités « eau » de Suez, ce qui en ferait le troisième opérateur mondial de la gestion de l'eau. L'autre inquiétude concerne la préservation des emplois d'ingénierie et des sièges. Cependant, Veolia soutient qu'en plus de conserver les deux masses salariales, l'entreprise continuera d'embaucher. est présenté, semble donc fournir toutes les garanties demandées : pas de situation de monopole, pas de suppressions d'emplois, et même l'obligation pour les parties prenantes de s'engager devant les parlementaires qui auront un droit de contrôle et de sanction sur les engagements non tenus. Pourtant, les élus locaux ne paraissent pas rassurés par les déclarations du président-directeur général de Veolia. En effet, la situation de concurrence actuelle leur permet d'obtenir des conditions de contractualisation favorables. Face à un groupe unique en situation de monopole, ce qui adviendrait si la fusion avec Suez aboutissait, les élus craignent d'être désavantagés et de voir leurs marges de manoeuvre fortement réduites.

concrètement à ces deux légitimes inquiétudes et intervenir dans ce dossier, afin de garantir à la fois une saine concurrence dans les territoires et le maintien des emplois existants ? La parole est à M. le ministre.

Après une alternance, au XX siècle, de périodes de fortes nationalisations et de périodes de privatisations, le portefeuille des entreprises à participation publique reste important. L'actualité récente montre cependant que l'État n'a pas toujours été efficace dans son rôle de protecteur du patrimoine économique et industriel de la France. On peut citer, sans être exhaustif, son rôle récent dans la cession de quelques-unes des principales entreprises cotées en Bourse : le Crédit lyonnais, les Autoroutes du Sud de la France (ASF), et, plus récemment, Alstom. Alors que le rôle de l'État consiste traditionnellement soit à accompagner le développement des filières stratégiques, soit à sauver les fleurons de l'industrie française, l'affaire Suez-Veolia exige que nous

dans l'affaire Carrefour. Il gagnerait d'autre part à réorienter tout ou partie de ses participations dans des domaines qui détermineront l'avenir des Français. Je pense bien sûr

Si l'État ne soutient pas le développement de semi-conducteurs chez STMicroelectronics ou ailleurs, il n'y aura pas de développement de semi-conducteurs, parce que l'investissement coûte trop cher et n'est pas rentable. Si nous ne soutenons pas massivement le développement de la filière hydrogène, aucun acteur privé ne pourra

que des entreprises veuillent conduire des stratégies de croissance et de développement, ou qu'un grand groupe veuille devenir le champion mondial des services dans le domaine de l'environnement : quoi de plus normal ? Toutefois, l'État actionnaire, l'État régulateur, l'État stratège, tel que vous venez encore de le redéfinir selon des orientations

mesure où l'État est le principal actionnaire d'Engie, il semble pour le moins ne pas s'être opposé au projet de Veolia. Il serait donc favorable à la création de ce géant mondial des services de l'environnement, dans des conditions de concurrence que vous nous avez précisées.

Monsieur le ministre, pourquoi accepte-t-on encore les OPA hostiles dans notre pays ? Elles ont pratiquement disparu aux États-Unis et dans les pays du nord de l'Europe. Hormis la fusion de la BNP et de Paribas en France, elles ont presque toujours échoué.

non seulement pour réconcilier les Français et l'entreprise, mais aussi pour reconquérir notre souveraineté nationale ? Peut-on imaginer une juridiction indépendante qui veille au respect de l'intérêt social de l'entreprise ? La parole

pour les élus locaux qui gèrent la ressource. Elle suscite, à ce titre, des préoccupations bien légitimes auxquelles l'État doit répondre, en prenant toutes ses responsabilités. Ces inquiétudes s'expriment notamment au sujet de la cession éventuelle par Veolia

Écrasé par les dettes, sera-t-il contraint de désinvestir presque la totalité de ce qu'il aura acheté ? Monsieur le ministre, quelles garanties avez-vous obtenues de la part de ce fonds d'investissement ? En effet, dans cette opération, nous savons ce que nous perdons-

monsieur le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat proposé par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, il me revient de conclure en tirant les enseignements des arguments formulés.

Plus largement, la question que pose cette affaire, comme d'autres affaires qui ont déjà défrayé la chronique, souvent quand il était trop tard pour les salariés et les territoires alors concernés, est de savoir quel rôle l'État français doit jouer auprès des entreprises françaises évoluant dans une économie de marché ouverte à la mondialisation, qu'il s'agisse pour l'État d'un patrimoine industriel dont il est pour partie détenteur, ou d'actifs considérés comme stratégiques sans qu'il en soit propriétaire. Quels sont aujourd'hui, hors situation de crise comme celle que nous vivons, les enjeux qui justifient que l'État prenne part au capital d'une entreprise- et à quel niveau ? -ou qu'il use de son influence pour sauver des actifs stratégiques ? De notre débat, il ressort que les enjeux à prendre en compte ont trait à l'emploi et à ses conséquences territoriales, à l'impact environnemental et à la soutenabilité du secteur économique concerné, à la compétitivité des entreprises dans un monde où les chaînes de valeur ont été décomposées à l'extrême, rendant souvent difficiles leurs relocalisations. Surplombant ces trois enjeux, la souveraineté nationale doit être en permanence notre boussole. Ce concept de souveraineté nationale doit être précisé par l'exécutif, débattu et évalué par le Parlement, peut-être dans le cadre d'une loi-cadre ou d'une loi d'orientation, L'affaire Veolia-Suez soulève à l'évidence des enjeux sociaux, économiques et environnementaux considérables pour notre pays. Or, depuis la sortie d'Engie du capital de Suez, qui a très vite suivi la non-reconduction de Mme Kocher et l'enclenchement de l'OPA hostile de Veolia, nous constatons un silence radio, ou presque, de la part du Gouvernement. Monsieur le ministre, quelle est la position du Gouvernement au sujet de ces deux grandes entreprises et de leurs actifs, que nous considérons comme stratégiques, compte tenu de leur importance sur les plans national et international ?

Quels sont les objectifs et les déterminants de la politique actionnariale et d'influence de l'État français en ce qui concerne les entreprises françaises à forts enjeux ? Quel sens donnez-vous au concept d'« État stratège » auquel, monsieur le ministre, vous vous référez si souvent ?

on le sait plus encore en 2021 qu'en 2019 -, qu'il s'agisse de santé, de climat, d'énergie, de défense, d'alimentation, et- je l'ajoute -de culture, tant la question démocratique en dépend de plus en plus par l'entremise du numérique. Dans chacun de ces domaines, et dans le cadre de politiques publiques de long terme, clairement explicitées et débattues, évaluées, le Parlement a un rôle éminent à jouer. Dans un monde en évolution rapide et profonde, au-delà de la médiatisation de quelques moments de crise à propos de telle ou telle entreprise en difficulté, ou du vote du compte d'affectation spéciale spéciale « Participations financières de l'État », dont nous ne cessons de dire, loi de finances après loi de finances, qu'il est très réducteur et peu clair, nous devons, nous parlementaires, engager avec les gouvernements un dialogue régulier, fondé sur l'intérêt général et national, autrement dit le temps long, et à l'aune des enjeux de l'emploi, de la compétitivité et de la soutenabilité que j'évoquais il y a quelques instants. Nous en sommes loin. Le Gouvernement, les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et cesser de s'abriter derrière le fait accompli ou le non-dit qui laisse place à toutes sortes d'interprétations. Il faut se le dire, il n'y aura pas de développement soutenable demain et, donc, de planète Terre vivable pour nos enfants si nous n'instaurons pas un autre rapport au temps, à la durée. Cela donne une responsabilité majeure aux États, censés être les garants du temps long. Le Gouvernement ne peut pas se comporter uniquement en banquier d'affaires. Si, dans l'opinion et chez les élus, les choix du Gouvernement semblent reposer sur des arrière-pensées non assumées, c'est l'intérêt national, qui a toujours une dimension locale, qui est amoindri. Or, dans une démocratie républicaine comme la nôtre, c'est inacceptable Il est grand temps que le gouvernement français donne une consistance à son concept d'« État stratège », qu'il discute et explicite sa politique actionnariale et sa politique publique d'influence économique. Une planification stratégique adaptée aux temps nouveaux devrait en résulter. Je ne crois pas me tromper en disant que la Chambre haute est prête à y apporter sa contribution. Ce débat de contrôle l'a amplement démontré. Je remercie d'ailleurs tous les groupes qui se sont exprimés.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, j'avais pris l'engagement devant vous, dès le 21 janvier, de poursuivre à vos côtés le travail normatif

En faisant prospérer l'initiative sénatoriale, le Gouvernement a fait le choix de saisir votre main tendue, mesdames, messieurs les sénateurs, pour dépasser les clivages sur un sujet qui nécessite notre mobilisation collective. Pour adopter les meilleures solutions que nous puissions apporter face à ces situations, il nous fallait conduire les réflexions avec hauteur de vue, nuance et discernement. Là aussi, c'est chose faite.

Trois dispositions fondamentales se sont clairement dégagées de nos échanges : la fixation d'un seuil d'âge à 15 ans, le renforcement de la répression de l'inceste et, enfin, l'allongement de la prescription en cas de pluralité des victimes. Nous y avons ajouté au cours des débats parlementaires à l'Assemblée nationale la prise en compte d'une réalité intolérable, la prostitution des plus jeunes, qui progresse malheureusement et qui doit être combattue sans relâche. Nous avons également pris en compte les remarques que le Sénat avait formulées en janvier dernier pour mieux réprimer tous les actes bucco-génitaux subis ou imposés. Ce sont donc au total cinq avancées incontestables qui figurent dans cette proposition de loi. Ces évolutions majeures sont de plus, je le crois, respectueuses de notre État de droit et, en particulier, des exigences constitutionnelles en matière de proportionnalité et d'égalité devant la loi pénale. C'est ainsi que, le 15 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté ces avancées historiques Je veux ainsi souligner la qualité des travaux menés par l'ensemble des parlementaires, en saluant en particulier l'implication tout à fait remarquable des rapporteures, Mme la députée Alexandra Louis et, bien sûr vous-même, madame la sénatrice Marie Mercier.

Permettez-moi également d'avoir un mot tout à fait particulier pour l'auteure de cette proposition de loi, la présidente Annick Billon dont l'engagement nous a, lui aussi, permis d'être réunis ici aujourd'hui. Je me désole, et je le dis de la manière la plus solennelle, de la campagne de désinformation, pour ne pas dire plus, dont vous avez pu faire l'objet, madame la sénatrice, au mépris total du travail conduit et des avancées réalisées. Je tiens donc, madame la sénatrice, dans cet hémicycle et en ce moment important, à vous adresser mes remerciements et à vous apporter mon plus chaleureux soutien. Je le sais et je l'ai déjà dit, si le sujet qui nous occupe aujourd'hui suscite les passions et sans doute beaucoup d'émotions légitimes, cette passion et ces émotions ne peuvent, en matière pénale, être nos seules guides. La passion et les émotions sont souvent mauvaises conseillères comme en témoignent les suggestions de toutes sortes, visent à renverser la charge de la preuve- pourquoi pas ? -, à prévoir des peines plus lourdes que pour le meurtre- pourquoi pas ? ou encore l'imprescriptibilité pour ces faits- pourquoi pas, là encore ? Je le dis solennellement, il est de notre devoir d'aborder cette question en responsabilité pour que la réponse juridique soit à la hauteur de l'attente des victimes que nous savons grande. Rien ne serait pire que de les décevoir en adoptant un dispositif bancal ou même contraire à notre Constitution. C'est pourquoi je me félicite que votre commission des lois ait voté en conscience ces avancées historiques tout en poursuivant le travail d'enrichissement du texte. Je ne doute d'ailleurs pas que la poursuite de nos débats nous permettra d'aboutir sur les tout derniers points restant en discussion. Le travail de pédagogie en direction de nos concitoyens est immense. C'est pourquoi il nous faut être concrets. Quels seront les effets de ce texte dans notre droit pénal ? Comment renforcera-t-il la protection des enfants face aux violences sexuelles commises par des adultes ? C'est à ces questions qu'il nous faut répondre clairement. Tout d'abord, aucun adulte ne pourra se prévaloir du consentement d'un mineur de 15 ans. Le texte prévoit d'ajouter de nouvelles définitions au crime de viol et au délit d'agression sexuelle, qui permettent d'exclure du débat judiciaire la question du consentement du mineur. Je l'ai dit, nos exigences constitutionnelles doivent être prises en compte. C'est pourquoi il nous faut garantir la proportionnalité de la répression, qui tend vers une criminalisation automatique de nombreuses situations. de l'écart d'âge de cinq ans qui permet de protéger les amours adolescentes. Parce que, qu'on le veuille ou non, nos adolescents ont une sexualité Parce que c'est la vie, parce que c'est leur vie ! Ne devenons pas les censeurs de leur vie sentimentale

l'instauration de cet écart d'âge n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de protéger des délinquants sexuels au bénéfice de leur jeune âge. Par ailleurs, tout en instaurant une loi pénale plus forte qui, en vertu de nos principes constitutionnels, ne s'appliquera que pour l'avenir, il nous faut maintenir un niveau très élevé de protection pour toutes les victimes de faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle. Ainsi, les dispositions issues de la loi de 2018 continueront de s'appliquer. Le viol et l'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sont évidemment maintenus. De même, le délit d'atteinte sexuelle ne sera pas supprimé, afin notamment de sanctionner des faits qui ne tomberont pas sous le coup des nouvelles qualifications, mais aussi de continuer de réprimer les faits commis avant la réforme. en effet pas envisageable de laisser sur le bord de la route les victimes passées d'abus sexuels commis par des majeurs, et d'adopter une réforme qui aurait pour conséquence d'amnistier les auteurs de ces actes. Autre avancée majeure, les viols les viols incestueux et les agressions sexuelles incestueuses seront désormais définis de manière autonome dans le code pénal et protégeront tous les mineurs le seuil d'âge est ici fixé à 18 ans. Les ascendants sont nécessairement visés par le viol incestueux et l'agression sexuelle incestueuse. L'oncle, la tante, le grand-oncle et la grand-tante, les neveux, nièces, frères et soeurs, les conjoints de ces derniers, les beaux-pères ou les belles-mères exerçant une autorité de fait ou de droit sur le mineur seront évidemment concernés. Pourquoi dès lors introduire la notion d'autorité de droit ou de fait dans le cadre des nouvelles incriminations incestueuses ? C'est parce que, en dehors des nous ne pouvons pas, automatiquement et sans individualisation, criminaliser la relation sexuelle en raison de liens de sang. Dans ces cas, il nous faut faire confiance au discernement et à l'appréciation des situations par les procureurs et par les juges. Vous les rencontrez régulièrement dans le cadre de vos travaux parlementaires, et vous connaissez leur engagement malgré la difficulté de leur mission : ils sont confrontés tous les jours à l'indicible à l'inaudible, et ils savent distinguer ce qui relève de la loi pénale. Je souligne avec force devant vous l'avancée réalisée en matière de relations incestueuses entre un majeur et un mineur puisque, désormais, les tribunaux n'auront plus à rechercher la violence, la contrainte, la menace ou encore la surprise. Autre évolution majeure, dans les situations où un même auteur réitère des crimes ou délits sexuels sur plusieurs victimes, je m'étais engagé à proposer un dispositif garantissant un traitement judiciaire égalitaire pour toutes les victimes. Les travaux normatifs nous ont conduits à instaurer un régime de prescription spécifique protégeant les mineurs. Le mécanisme de prescription prolongée, qui permet de faire bénéficier toutes les victimes de la prescription la plus longue,

même si le dernier crime n'est finalement pas poursuivi faute de preuves, ou s'il fait l'objet d'un acquittement, les autres crimes révélés grâce à ce dernier crime pourront tout de même être jugés. je l'ai évoqué au début de mon propos, la situation des mineurs victimes de prostitution est bien prise en compte. Désormais, grâce aux nouvelles incriminations, tout majeur de 18 ans

en incluant, non seulement la relation sexuelle rémunérée, mais également la promesse de rémunération, la fourniture d'un avantage en nature ou la promesse d'un tel avantage. Cette disposition contribue à renforcer véritablement la protection de nos mineurs. C'est dans ce même esprit que votre commission a autorisé l'extension du nouveau délit de « sextorsion » à tous les mineurs de 18 ans. Vous le voyez,

sur de nombreux aspects de la protection que nous devons à nos mineurs face aux violences sexuelles qu'ils subissent. L'ambition historique qu'il porte nous permettra de dire solennellement aux victimes : il y aura un « avant »

il y a exactement dix jours, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi dont le titre a changé, puisqu'elle vise désormais « à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

Ces votes successifs montrent que le texte répond à une attente : dans leur grande majorité, nos concitoyens demandent un renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par les adultes. L'objectif principal est qu'il ne soit plus nécessaire de s'interroger sur la question du consentement du jeune mineur eu égard à son manque de maturité et de discernement. Rappelons-nous le « un homme ça s'empêche » de Camus. Il est effectivement de la responsabilité de l'adulte de respecter des limites pour préserver l'intégrité physique et psychique des enfants et des adolescents. Je crois que nous en sommes tous d'accord. En première lecture, nous avions estimé que la création d'une infraction autonome de crime sexuel sur mineur, avec un seuil d'âge fixé à 13 ans, répondait à nos objectifs.

Il nous faut cependant reconnaître que le choix d'un seuil d'âge à 13 ans, même s'il s'appuie sur de solides justifications, a pu être mal compris et parfois perçu comme un recul par rapport au seuil de 15 ans qui vaut pour le délit d'atteinte sexuelle.

Avec l'appui de la Chancellerie, l'Assemblée nationale a imaginé une solution différente, qui tient compte de nos préoccupations, tout en étant mieux comprise par les associations de protection de l'enfance, comme les auditions auxquelles j'ai procédé me l'ont montré. Dans le texte qui nous est transmis, le seuil d'âge est fixé à 15 ans, mais il est assorti d'un écart d'âge de cinq ans entre l'auteur des faits et la victime : de cette manière, les relations consenties entre un mineur âgé d'un peu moins de 15 ans et un tout jeune majeur, relations qui ont d'ailleurs pu débuter alors que les deux partenaires étaient mineurs, ne seront pas C'est le terme « automatiquement » qui importe ici. Le choix de créer une infraction autonome avait également suscité des réserves, certains lui reprochant d'évacuer la dimension violente du passage à l'acte, qui serait mieux prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression sexuelle. Sur ce point également, l'Assemblée nationale a fait preuve d'esprit de synthèse en décidant de qualifier de viol la nouvelle infraction sexuelle Je tiens à dire que certaines infractions prévues par le code pénal renvoient à plusieurs définitions. C'est le cas par exemple pour le harcèlement sexuel, qui suppose en principe la commission d'actes répétés, mais qui peut aussi être constitué si un acte unique particulièrement grave a été commis. Tel serait désormais le cas aussi pour le crime de viol : à la définition classique, qui suppose un élément de contrainte, de menace, de violence ou de surprise s'ajouterait une nouvelle définition, qui ne sera applicable que si la victime est un mineur de 15 ans. Concernant la définition du viol, je signale que l'Assemblée nationale a conservé la mesure que le Sénat avait adoptée, sur l'initiative de nos collègues Esther Benbassa et Laurence Rossignol, qui tend à l'élargir aux actes bucco-génitaux. Il s'agit d'une avancée importante, ces actes pouvant être tout aussi traumatisants pour la victime qu'une pénétration sexuelle. Sur la question de l'inceste, le texte renforce la protection de tous les mineurs jusqu'à 18 ans en introduisant deux nouvelles infractions de crime incestueux et d'agression sexuelle qui seront constituées si les faits sont commis par un ascendant ou par un membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Par membre de la famille, il faut entendre les frères et soeurs, les oncles et tantes, les neveux et nièces, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires de PACS. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter à cette liste les grands-oncles et les grands-tantes. Je sais que l'exigence d'une autorité de droit ou de fait a pu susciter des interrogations. Après réflexion, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il s'agit d'un critère essentiel à la cohérence d'ensemble du dispositif : en l'absence d'une relation d'autorité, comment distinguer en effet l'auteur des faits de la victime ? Certains diront que le partenaire majeur est forcément coupable, mais cette affirmation ne résiste pas à un examen objectif de la diversité des situations que l'on peut rencontrer sur le terrain. sur le terrain. Dans une famille, un fils de 17 ans peut fort bien avoir l'ascendant sur le reste de la fratrie, y compris sur sa soeur de 18 ans et demi. Si le père est absent, il arrive même parfois que le fils aîné se comporte quasiment en chef de famille. En cas de relation incestueuse, il convient donc d'examiner chaque situation au cas par cas- c'est le rôle du juge -, afin de déterminer qui a imposé l'acte sexuel, sans quoi nous nous exposerions à un risque élevé d'erreurs judiciaires. J'en arrive à la question un peu complexe de la prescription pour vous indiquer que l'Assemblée nationale a maintenu l'allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation d'infraction sur mineur, que le Sénat avait adopté, en le recentrant sur les crimes et délits sexuels, ce qui est cohérent avec l'objet du texte. En ce qui concerne la prescription des crimes et délits sexuels eux-mêmes, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un double mécanisme. Le premier s'inspire de celui que le Sénat a introduit. Il aurait pour effet de prolonger le délai de prescription d'un crime ou délit sexuel sur mineur si l'auteur commet un autre crime ou délit sexuel sur un autre mineur. Le deuxième mécanisme s'inspire de la notion de connexité : un acte interruptif de prescription, une audition par exemple, interromprait la prescription, non seulement dans l'affaire considérée, mais également dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée au même auteur la commission d'un autre crime ou délit sexuel sur mineur. Avec ces deux dispositifs, toutes les victimes pourront comparaître comme telles devant la cour d'assises, alors que les victimes les plus « anciennes » sont seulement entendues en tant que témoins Je sais que le garde des sceaux, fort de sa longue expérience d'avocat pénaliste, est sensible à cette évolution, que notre commission a approuvée. J'évoquerai enfin les autres dispositions qui figurent dans le texte. Tout d'abord, l'Assemblée nationale a conservé les mesures à caractère préventif que nous avions adoptées sur l'initiative de Michel Savin et de Valérie Boyer. Elles tendent à élargir la liste des infractions entraînant une inscription incitent les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec un mineur. L'Assemblée nationale a enrichi le texte sur l'initiative de la rapporteure Alexandra Louis de manière à mieux réprimer des phénomènes nouveaux apparus sur internet et, je dois le dire, très inquiétants, par lesquels des majeurs demandent à des mineurs d'accomplir des actes obscènes devant une caméra, leur demandant de se filmer à un, à deux, à trois, puis de leur envoyer les images. Parfois qualifiés de « sextorsion », ces agissements peuvent ouvrir la voie à un véritable chantage exercé sur le mineur pour l'amener à accomplir des actes de plus en plus avilissants. Je vous propose d'approuver ces dispositions nouvelles, afin que la loi pénale exprime clairement notre refus de ce type de comportement. Au total, le texte qui vous est soumis renforce vraiment la protection des mineurs au prix, il est vrai, d'une plus grande complexité des règles de droit applicables. Un travail de pédagogie devra être mené par la Chancellerie auprès des juridictions et je souhaite que nous puissions, après l'adoption de ce texte, stabiliser les règles applicables aux infractions sexuelles sur mineurs afin que les professionnels du droit aient le temps de se les approprier. Ce texte donne des outils au juge avec le but, que nous partageons tous, de diminuer le nombre de décisions de classement sans suite. Le regard du juge évolue aussi avec la société. La commission vous propose de préserver les grands équilibres du texte. Certes, il n'est pas parfait, mais je suis convaincue qu'il marquera une étape importante dans nos politiques de sauvegarde de l'enfance. Il faudra bien sûr l'accompagner de mesures de prévention et d'éducation dans les écoles, dans les milieux sportifs, dans les associations et, surtout, dans les familles. Ces mesures ne relèvent pas du domaine de la loi, mais elles sont décisives pour préserver les enfants et les adolescents contre les violences sexuelles. Je suis également convaincue qu'il ne suffit pas de changer la loi : ce sont aussi les mentalités qui doivent évoluer. Vraiment, nous devons

À l'exception de quelques soixante-huitards qui ne se sont rien interdit, même pas les rapports sexuels avec des mineurs, et qui continuent à bénéficier d'une certaine et nauséabonde bienveillance médiatique, voici un texte avec lequel l'ensemble des Français seront d'accord : protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Cependant, nous en avons fait l'expérience, le Sénat a été pris pour cible à l'issue de la première lecture par une certaine presse qui a relayé à grand renfort de titres raccourcis les intentions contraires à celles que nous avions souhaité donner à ce texte. Quel était le but de cette campagne, sinon de désinformation, à tout le moins de déformation ? Déstabiliser le Sénat en sa qualité de contre-pouvoir démocratique ? Décrédibiliser l'initiative parlementaire des élus représentant les territoires ? Ce qui est certain, c'est que les Français sont à cran ; en témoigne l'ampleur prise dans l'opinion par le vote à l'unanimité de ce texte. Je veux donc dire ici, mes chers collègues, pour que nos conclusions soient claires, je veux surtout le dire à ceux qui suivent nos travaux, aux victimes qui attendent beaucoup de la protection de la loi, ainsi qu'aux parents qui craignent pour la sécurité de leurs enfants : non, le Sénat n'a pas abaissé la majorité sexuelle à 13 ans oui, le Sénat votera ce texte, je l'espère à l'unanimité, et nous continuerons de faire évoluer notre droit pour que les personnes se rendant coupables de viol, de viol sur mineur, de viol incestueux, de harcèlement, d'agression, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle ou d'acte justifiant toute autre circonstance aggravante soient poursuivies, et sévèrement punies. Et, pour cela, il convient de rappeler que le coeur de cette proposition de loi est la création d'un nouveau crime sexuel sur mineur de 15 ans. Mais elle permet aussi, après évolutions, l'élargissement de la définition du viol et du crime sexuel sur mineur l'allongement des délais de prescription. Elle crée aussi deux nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse. Enfin, elle élargit la liste des infractions entraînant l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Alors, mes chers collègues, je vous appelle à être consciencieux : ne manquons pas de cohérence et de lisibilité. Il faut une loi compréhensible par tous, qui ne soit pas interprétable par tous les complices de l'abject qui essaient encore de salir, de blesser, de violer psychologiquement par les écrits odieux qu'ils ont encore l'occasion de publier. Sachons rédiger un interdit clair autant que nous devons voter des peines sévères, exemplaires, à la hauteur de l'ignominie que constituent les actes pédocriminels, à la hauteur de l'attente des victimes et de leur famille.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous nous réunissons, de nouveau, aujourd'hui pour garantir à nos enfants une meilleure protection contre les violences sexuelles. Depuis trop longtemps, nous constatons le décalage entre la réalité des violences faites aux enfants et le regard que portent les institutions, mais aussi une partie de la société, sur ces violences. Longtemps, nous n'avons proposé aux victimes qu'une alternative inadéquate : soit le silence, soit des réponses à la fois incomplètes en matière d'accompagnement et complexes sur le plan judiciaire. C'est pourquoi je me réjouis que des étapes importantes aient été franchies au cours de ces dernières années. Désormais, bien plus qu'hier, on écoute les victimes, on les croit, on les aide. Toutefois, si la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a déjà permis des avancées majeures, il nous faut aller plus loin encore pour que les choses soient désormais claires pour toutes et tous : on ne touche pas à l'innocence des enfants La proposition de loi déposée par notre collègue Annick Billon s'inscrit dans l'esprit de très nombreux travaux parlementaires déjà menés avec engagement au Sénat et tente de répondre à un terrifiant constat 80 % environ des violences commencent avant 18 ans, la première agression survenant en moyenne à l'âge de 9 ans. Dans plus de 90 % des cas, elles sont commises par des proches. Aussi, je me félicite que l'Assemblée nationale ait souhaité contribuer à améliorer la protection des mineurs contre ces violences. Notre commission a travaillé à parfaire les équilibres qui ont pu être trouvés : il était indispensable de préserver celui de l'échelle des peines il était aussi nécessaire de procéder à plusieurs ajustements, notamment en créant de nouvelles circonstances aggravantes. Ce texte durcit également les sanctions de l'inceste et prévoit l'interruption de plusieurs délais de prescription. Ce faisant, la proposition de loi que nous examinons atteint deux objectifs : elle améliore la protection des victimes ; elle envoie, ensuite, un message clair et fort en rappelant à tous les adultes la nécessité de protéger les enfants. Si les mineurs de 15 ans sont particulièrement vulnérables, nous considérons que les mineurs, dans leur ensemble, sont des personnes vulnérables à qui nous devons une protection accrue. Nous nous réjouissons donc que la rédaction des nouveaux délits de « sextorsion » sur internet ait été modifiée et protège à présent tous les mineurs. Avant de conclure, je tiens à remercier Annick Billon, auteure de cette proposition de loi qui consacre un combat de plusieurs années, mais aussi Marie Mercier, pour son engagement sur ce sujet et la qualité de ses travaux. Enfin, j'ai une pensée pour toutes les victimes, dont certaines nous écoutent peut-être aujourd'hui. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants soutient cette proposition de loi, en espérant que, après les nombreuses discussions qui ont déjà eu lieu sur ce sujet au sein de notre assemblée, ce texte recueillera un accord transpartisan et que, surtout,

la deuxième lecture de cette proposition de loi que nous devons d'abord, il convient de le rappeler, à notre chère collègue Annick Billon, que je salue, est la démonstration parfaite des progrès sociétaux qui peuvent naître d'un travail commun et transpartisan entre les deux assemblées. L'urgence était indéniable ; il convenait de faire évoluer la loi pour mieux protéger les quelque 160 000 mineurs qui, selon les estimations, subissent chaque année en France des violences sexuelles. Il convenait aussi d'apporter une réponse juste à la libération de la parole des victimes d'inceste, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MeeTooInceste, mais aussi avec les récentes affaires révélées dans les médias

que nous saluons, d'inscrire ce texte à leur ordre du jour, de l'amender positivement pour aboutir à cette version qui nous convient, à mon groupe et à moi-même. Parmi les nouveautés issues de la navette parlementaire, la réécriture de l'article 1, qui vise à sanctionner tout acte sexuel commis par un majeur sur une personne mineure de 15 ans, est une amélioration significative. Désormais, la pénétration ou l'acte bucco-génital commis par un majeur sur une personne de moins de 15 ans sera qualifié de viol. Le relèvement de ce seuil de 13 ans à 15 ans était une demande de certaines d'entre nous. D'ailleurs, toutes les sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, auquel j'appartiens, avaient cosigné, en première lecture, l'amendement déposé en ce sens par Mme Laurence Rossignol. Nous nous satisfaisons également du renforcement du dispositif d'interruption du délai de prescription en cas de commission d'un même crime par un même auteur à l'endroit d'autres mineurs. Nous nous félicitons en outre de ce que le rapport bucco-génital soit reconnu comme viol au même titre que la pénétration sexuelle. Mon groupe avait notamment pris l'initiative de déposer un amendement qui allait dans ce sens. Enfin, et surtout, nous nous réjouissons que la France ait finalement le courage de reconnaître dans son droit l'inceste comme crime en soi.

que nous ne pouvions plus ignorer, quand près de 6,7 millions de Françaises et Français en auraient été victimes, selon une étude menée par l'association Face à l'inceste. Il revient maintenant à l'État de se pencher plus encore sur le sujet et de produire régulièrement des données officielles précises qui permettront de prendre toute l'ampleur de la réalité des violences sexuelles commises sur les personnes mineures. Cette proposition de loi nous semble protectrice ; elle constitue une réelle avancée sociétale. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte. La

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, nous examinons aujourd'hui, en deuxième lecture, la proposition de loi de notre collègue Annick Billon visant à mieux protéger les mineurs des crimes sexuels. Le 21 janvier dernier, nous adoptions à l'unanimité ce texte, qui prévoyait initialement d'introduire au sein du code pénal un nouveau crime autonome, puni de vingt ans de réclusion criminelle et caractérisé par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit [ ...], commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans Pour la première fois, au-delà des clivages qui traversent notre assemblée, nous inscrivions dans la loi un seuil d'âge de non-consentement, 13 ans à l'origine, afin de criminaliser tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant. Lors de a fait l'objet de modifications importantes que nous tenons à saluer. Nous avons tous à l'esprit les innombrables témoignages, de personnalités publiques ou d'anonymes, qui ont contribué à lever le tabou autour de l'inceste et à enfin libérer la parole des victimes. En y intégrant un crime de viol incestueux et un délit d'agression sexuelle incestueuse, ce texte met fin aux lacunes de la loi sur ces actes et à notre aveuglement collectif sur ce que vivent 10 % des enfants, bien souvent livrés à eux-mêmes et contraints au silence. En vertu de cette proposition de loi, l'inceste constitue désormais une infraction spécifique, assortie de sanctions propres, et non plus uniquement une surqualification pénale. Tous les mineurs jusqu'à 18 ans seraient protégés par ces nouvelles dispositions. Je m'en réjouis, car, non, il n'existe pas d'inceste consenti ou « heureux » ; il s'agit toujours d'un calvaire qui hante les victimes, parfois tout au long de leur vie. L'article 1, au coeur de cette proposition de loi, a donc été récrit. Un interdit est désormais posé à 15 ans, ce qui conduit à ne plus interroger le consentement du mineur en dessous de cet âge. Il s'agit ici d'une avancée majeure unanimement saluée. Ce texte pose un principe clair : en dessous de 15 ans, c'est non Il était toutefois nécessaire d'apporter un aménagement pour éviter de criminaliser les amours adolescentes, qui existent et, nous le savons, continueront d'exister dans notre société. Ce texte prévoit donc désormais quatre infractions qui ne nécessitent pas d'établir une violence, contrainte, menace ou surprise, allant ainsi dans le sens d'une meilleure protection des mineurs. Cet enrichissement, salué par tous, démontre la capacité de nos assemblées à surmonter ses oppositions lorsque l'intérêt général, et surtout celui de nos enfants, est en jeu. Nous saluons également la création, par voie d'amendement, du délit de « sextorsion », lorsqu'un majeur incite un mineur, sur les réseaux sociaux, à commettre un acte de nature sexuelle sur lui-même ou sur un tiers, y compris si cette provocation n'est pas suivie. Ce nouveau délit tend à prendre en compte l'évolution des rapports et l'appétence des jeunes, parfois des très jeunes, pour les réseaux sociaux. Grâce à ce délit de « sextorsion », le droit s'adapte à l'apparition de nouvelles formes de criminalité en ligne dont les mineurs sont victimes et qui conduisent bien souvent à des drames. Enfin, cette proposition de loi crée un mécanisme de prescription prolongée dans le cadre de crimes sériels. Sur proposition du garde des sceaux, un deuxième mécanisme a été introduit visant à ce qu'un acte interruptif de prescription puisse prendre effet non seulement seulement dans l'affaire considérée, mais également dans les autres procédures dans lesquelles serait reprochée, au même auteur, la commission d'un autre crime ou délit sur mineur. À titre personnel, je souhaite que nous ayons un débat sur l'existence même du délai de prescription pour les actes sexuels commis sur des mineurs. Pour conclure, je tiens à saluer le travail de notre collègue Annick Billon. L'adoption, je l'espère, de ce texte, aboutira à une meilleure protection des mineurs. Je remercie également la rapporteure Marie Mercier, dont les amendements ont permis de renforcer juridiquement cette remercie enfin le Gouvernement pour les concertations qu'il avait annoncées dans notre hémicycle et qui ont été menées pour faire évoluer ce texte. Pour ces raisons, le groupe RDPI votera cette proposition de loi.

d'apporter tout le soutien du groupe du RDSE à la présidente Carole Delga et à nos collègues conseillers régionaux d'Occitanie, qui ont subi cet après-midi, durant leur séance plénière à Toulouse, une violente intrusion d'extrémistes de l'Action française. Nous condamnons avec fermeté cette atteinte au fonctionnement d'une institution de notre République et, symboliquement, à notre démocratie. J'en viens au texte. Au mois de janvier dernier, le Sénat adoptait à l'unanimité cette proposition de loi visant à instituer une nouvelle incrimination pénale de crime sexuel sur mineur. Le groupe du RDSE et moi-même tenons à redire tout notre soutien à l'auteure de cette proposition de loi, Annick Billon, victime, à l'époque, d'une polémique et d'un traitement médiatique injuste et regrettable. Elle aura eu le mérite de remettre l'ouvrage sur le métier et d'engager de nouveau le Parlement dans un travail visant, d'une part, à proposer un meilleur dispositif de condamnation des auteurs de violences sexuelles sur mineur et, d'autre part, à enfin pouvoir instituer une véritable condamnation pénale de l'inceste. Désormais, ce nouveau texte comprend ce que beaucoup avaient appelé de leurs voeux, à savoir la condamnation des crimes sexuels sur les mineurs de 15 ans. Il faut le redire : en aucun cas, le Sénat n'avait adopté en première lecture une loi autorisant les relations sexuelles entre un majeur et un mineur à partir de 13 ans. Au contraire, le dispositif voté venait renforcer la protection des enfants. Ainsi, grâce à l'apport de l'Assemblée nationale, ce renforcement bénéficiera également aux enfants de 13 ans à 15 ans. Jusqu'à cet âge, il ne sera donc plus nécessaire de rechercher l'existence d'un consentement chez l'enfant qui justifierait l'acte de l'adulte. Sur la question de l'inceste, ensuite, en 2019,

Certes, lors de nos débats en première lecture, nous avions buté sur des difficultés d'ordre juridique, quand bien même la condamnation de l'inceste dans son principe ne soulevait pas de difficultés. Mais l'Assemblée nationale a pu poursuivre nos travaux et proposer un texte satisfaisant, même s'il n'est pas parfait, qui pourrait mettre fin à une anomalie qui existe depuis trop longtemps dans notre droit : l'absence d'infraction spécifique visant l'inceste. Parmi les autres innovations apportées au texte initial, il faut aussi souligner celle qui vise à sanctionner plus durement les prédateurs qui utilisent internet pour forcer les mineurs à accomplir sur eux-mêmes les actes les plus dégradants. Il s'agit ici aussi d'un fléau qui peut briser durablement la vie de certains enfants et auquel nous devons aussi apporter une réponse pénale. Ce point tient particulièrement à coeur à notre rapporteure, que je salue, et que je remercie du travail qu'elle Enfin, nous observons une actualité médiatique qui révèle de plus en plus régulièrement des affaires de violences sexuelles sur mineurs. Face à ces faits, nous devons apprendre à mieux recevoir la parole des enfants victimes, à faciliter leur accompagnement dans sa dimension judiciaire, certes, mais également dans sa dimension humaine et sociale. Il faut qu'il n'y ait aucun doute pour les victimes de ces abus qu'elles seront soutenues par notre nation. Dans cette perspective, j'aimerais me réjouir que, malgré certains événements, la commission indépendante sur les violences sexuelles sur mineur ait été maintenue. Il a fallu qu'elle soit recomposée, mais il est certain que ses travaux contribueront à nous éclairer sur un sujet complexe et difficile, mais également fondamental. En conclusion, je reprendrai l'avertissement de l'un des nouveaux membres de la commission, le thérapeute et écrivain Jean-Paul Mugnier. Il explique : « Ne détournons pas de nouveau notre regard de celui des enfants, qui, désespérés, tentent de nous faire savoir le mal dont ils sont les victimes. » Il écrivait ces mots en 1999, voilà plus de vingt ans. Cela doit nous faire réaliser combien il aura fallu de temps

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, après notre travail en première lecture sur la proposition de loi présentée par notre collègue Annick Billon, que je tiens une nouvelle fois à remercier, ce nouveau rendez-vous pour parfaire la protection des mineurs contre les crimes et délits sexuels était très attendu, d'autant que le travail du Sénat avait fait naître une polémique injustifiée dans les médias, du fait d'une interprétation erronée. Les tabous sont levés, la cause des enfants victimes de ces violences sexuelles brise, fort justement, le mur du silence. C'est notamment grâce aux associations de protection de l'enfance et aux nombreuses victimes qui ont continué à se battre. Elles ont démontré, à juste titre, la nécessité de faire évoluer notre droit pour une loi plus claire posant un interdit sans ambiguïté et, surtout, sans avoir à interroger le consentement prétendu de la victime. L'interdit est clairement posé ici aucun adulte n'a le droit d'avoir des rapports sexuels avec un ou une enfant ; fixation d'un seuil de 15 ans, reporté à 18 ans pour l'inceste. C'est une bonne chose, mais, malheureusement, ce seuil est assorti, en dehors de l'inceste, d'une condition d'écart d'âge de cinq ans pour prendre en compte la « clause de Roméo et Juliette Même si nous avons bien compris que cet écart n'aurait plus lieu d'être dès lors qu'un des éléments classiques du viol serait présent, nous craignons que cette rédaction ne limite véritablement la portée de cette mesure et ne nous fasse retomber dans les mêmes débats autour du consentement. En effet, 65 % des violeurs de mineur ont entre 18 ans et 24 ans et certaines victimes de 14 ans, par exemple, seront par conséquent moins bien protégées. Nous devons y réfléchir. Par ailleurs, en première lecture, mon groupe avait déposé un amendement pour compléter la définition du viol et instaurer une présomption de contrainte, estimant que la création d'une infraction autonome sans jamais utiliser le mot « viol » posait problème. L'ajout par l'Assemblée nationale de ce terme, et parce que les mots ont un sens, nous convient. Si nous nous réjouissons que les débats à l'Assemblée nationale aient permis de considérer l'inceste non plus comme une circonstance aggravante, mais bien comme une infraction à part entière, vous proposez en quelque sorte de le « conditionnaliser » à la notion d'autorité, de droit ou de fait. N'est-ce pas une porte ouverte pour les agresseurs qui ne sont pas dans une situation d'autorité, de droit ou de fait ? En revanche, notre groupe soutient sans réserve le nouveau délit créé pour des faits de « sextorsion », qui va plus loin que la corruption de mineur en s'adaptant à la réalité d'aujourd'hui, à savoir le tout-numérique et l'utilisation d'internet. Enfin, nous soutenons le mécanisme nouveau de prescription glissante pour permettre la prolongation du délai de prescription en cas de nouvelles infractions, tout en entendant les réserves du Syndicat de la magistrature sur l'imprescriptibilité de fait. définitive, ce texte crée de nouvelles infractions allant du crime au délit pour essayer de couvrir un champ très large. Mais attention ! Attention à la complexité de tous ces dispositifs : le principe de lisibilité de la loi est ainsi sérieusement écorné, et il nous faut bien en mesurer les conséquences. Mes chers collègues, ce texte est important : il est le fruit d'un long travail, notamment celui de Marie Mercier, que je veux saluer, d'un travail collectif pour améliorer ces définitions du viol et de l'agression sexuelle, qui ne pouvaient être les mêmes quand on parle de mineur. Je regrette néanmoins que, tout en apportant de belles avancées, il affaiblisse parfois la portée du texte initial, en créant des dérogations. De même, je m'interroge sur la façon dont vont se avec le travail sur l'inceste de la commission indépendante coprésidée par Édouard Durand ou avec celui du groupe de travail contre la prostitution des mineurs. Mes chers collègues, au-delà du répressif et du suivi des auteurs, nous devons nous interroger sur le rapport de notre société à ce phénomène des violences faites aux enfants, agir sur les mentalités par l'éducation, la déconstruction des stéréotypes sexistes. C'est une urgence. Nous devons également prendre le temps d'évaluer les politiques qui sont mises en place, judiciaires, mais pas seulement : je pense notamment à la pratique de la correctionnalisation ou encore à l'accueil, à l'accompagnement des victimes, à la formation des professionnels. Comment ignorer que les brigades locales de protection des mineurs sont en souffrance s'agissant des effectifs et des moyens ? En attendant, cette loi est une étape importante dans la lutte pour protéger les enfants contre les délits et crimes sexuels, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La parole

nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour examiner ma proposition de loi, modifiée, qui intègre désormais les crimes et délits incestueux. Le 21 janvier dernier, le Sénat inscrivait pour la première fois dans la loi un seuil d'âge de non-consentement à 13 ans. L'inadaptation des critères du viol et l'impossibilité pour un enfant de consentir à une relation sexuelle avec un adulte étaient enfin reconnues. La Haute Assemblée a ainsi ouvert la voie en adoptant ce texte à l'unanimité. Parce qu'il est difficile d'obtenir un tel consensus, ce vote témoigne de la capacité du Sénat à s'emparer d'un sujet trop longtemps passé sous silence. Ce texte, discuté à l'Assemblée nationale le 15 mars dernier, revient enrichi et modifié grâce à un travail de coconstruction entre le Parlement et le garde des sceaux. Je souhaite à ce titre remercier tous ceux qui ont contribué à son amélioration : Mme la rapporteure Marie Mercier, la commission des lois du Sénat, la rapporteure de l'Assemblée nationale, Mme Alexandra Louis, les députés, le Gouvernement et, enfin, le groupe Union Centriste et son président Hervé Marseille, qui a pris le risque d'inscrire à notre ordre du jour cette proposition de loi à l'autonome dernier, à un moment où où ce sujet ne faisait pas consensus. Très bien ! La commission des lois du Sénat, par la voix de sa rapporteure, a souhaité retoucher le texte issu de l'Assemblée nationale. Ses amendements ont pour but non pas de remettre en cause les grands équilibres trouvés, mais de nous assurer de sa cohérence juridique. Il y va de la protection des victimes. Nous nous devons d'apporter une réponse pénale ferme et adaptée à ce qui relève d'un phénomène de masse : 60 % des victimes de violences sexuelles sont des enfants. Et, alors que les victimes de viol sont au nombre de 300 000 chaque année, seuls 0,3 % des violeurs sont condamnés. Pendant trop longtemps, nous avons fait preuve d'impuissance, voire d'incurie, dans le traitement de ce fléau. Sur les violences sexuelles sur mineurs, spécifiquement dans le cadre intrafamilial, nous avons été frappés de cécité. Et pour cause, nos sociétés ont érigé depuis plusieurs siècles le foyer en sanctuaire : difficile, alors, d'appréhender les atrocités étouffées qui peuvent se jouer dans le huis clos familial. Il aura fallu plusieurs étapes, plusieurs lois, plusieurs ouvrages, plusieurs témoignages pour que la parole se libère massivement, mais aussi et surtout pour que l'on entende enfin la voix de ces enfants. À présent, ces agissements seront qualifiés et reconnus dans le code pénal comme des infractions spécifiques. Celles-ci porteront les noms de « viol sur mineur » », « viol incestueux », « agression sexuelle sur mineur » et « agression sexuelle incestueuse Nos collègues députés ont introduit des dispositions nouvelles, sur l'inceste, tout d'abord. Désormais, l'inceste est reconnu comme une infraction spécifique et puni à hauteur de sa gravité lorsque la victime est mineure. Les députés ont également opté pour le relèvement de 13 ans à 15 ans du seuil à partir duquel tout rapport sexuel entre une personne majeure et un mineur est un crime.

Nous sommes animés par un objectif commun, celui de mieux protéger nos enfants face aux agresseurs sexuels. Et, si je reconnais la portée symbolique de ce seuil fixé à 15 ans, je reste cependant convaincue que le dispositif initial avait pour lui l'avantage de la clarté et celui de la sécurité juridique et constitutionnelle. Ce dispositif avait malheureusement été mal compris au moment de son adoption, et des interprétations erronées et abusives avaient prospéré, déduisant à tort que le Sénat avait abaissé l'âge du consentement à 13 ans. L'Assemblée nationale a également précisé l'apport du Sénat en matière de prescription.

Ce texte apporte des avancées majeures et attendues, car il entérine un virage décisif dans la manière d'appréhender les violences sexuelles sur les mineurs. À présent, un enfant ne sera plus jamais considéré comme complice ou complaisant à l'égard des actes sexuels qu'un adulte commet sur lui. Ce changement de paradigme est fondamental dans la reconstruction future des enfants : en reconnaissant intégralement leur qualité de victime, la justice les libérera du poids d'une culpabilité éprouvée à tort. chers collègues, en 2018, à l'occasion du vote sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, j'avais, devant cette assemblée, posé la question suivante : les dispositions proposées permettront-elles réellement de protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et d'en finir avec l'impunité des agresseurs ? Je n'en étais pas convaincue. Aujourd'hui, je me félicite de ce que vous permettiez à cette proposition de loi d'atteindre pleinement cet objectif. C'est une étape majeure qui est franchie. La prévention et la formation doivent désormais s'ajouter au droit

un hommage aux victimes qui ont eu l'énergie et le courage de parler, un hommage aux associations qui se sont battues depuis tant d'années, un hommage aux parlementaires, Annick Billon, mais aussi Laurence Rossignol, Michelle Meunier, Isabelle Santiago.

a fait que la société a bougé, et elle a fait que nous, parlementaires engagées depuis longtemps sur ces sujets, avons pu trouver du soutien pour faire avancer cette cause.

Nous pouvons voir les choses positivement : il a donc fallu que les semaines passent pour qu'en définitive chacun se rende à la raison et décide de soutenir les propositions qui furent les nôtres. Soyons donc optimistes, ou plutôt positifs, et notons les progrès accomplis ; ils sont incontestables. Un grand nombre de mesures de ce texte doivent être retenues et saluées.

permet de qualifier d'« amours adolescentes » les relations sexuelles entre un jeune de 19 ans et un jeune de 14 ans.

La deuxième difficulté que nous constatons tient à la notion d'autorité de droit ou de fait. Je pense qu'il y a une confusion sur ce sujet : l'inceste n'est pas un crime de pouvoir ; l'inceste est un interdit anthropologique.

soient écartés, nous envisageons de ne pas voter pour ce texte, car nous souhaitons qu'il progresse encore, dans le cadre des échanges au sein de la commission mixte paritaire

nous sommes réunis une nouvelle fois cet après-midi pour étudier la proposition de loi de notre collègue Annick Billon, après son examen en première lecture à l'Assemblée nationale. Nul besoin de souligner ici l'importance du sujet, tant l'actualité nous rappelle, presque chaque semaine, que des enfants ont souffert, souffrent, et risquent de souffrir encore si rien ne change. C'est l'honneur du Sénat que d'avoir mis à l'agenda politique, par le biais de cette proposition de loi, la question d'une révision de notre droit en matière de crimes sexuels sur mineurs. Nous en avons collectivement fait le constat : si la dernière réforme date de 2018, elle ne résout pour autant pas l'ensemble des problèmes que la libération de la parole des victimes et celle, non moins importante, de l'écoute qui leur est accordée ont contribué à mettre au coeur des priorités politiques. Les débats en première lecture ont été riches et, me semble-t-il, la navette parlementaire a rempli son office. La preuve en est que le Gouvernement a décidé de reprendre le texte issu du Sénat pour faire aboutir la réforme- il nous faut le souligner. Nous le savons : l'Assemblée nationale a décidé de fixer le seuil de non-consentement à un rapport sexuel avec un mineur à 15 ans, contre 13 ans proposés par le Sénat. Nous ne nous opposerons pas à ce nouveau seuil, même si les retours du terrain nous font craindre une application juridique plus complexe pour les professionnels concernés.

Nous avons jugé, en conscience, qu'une telle censure aurait constitué un signal extrêmement déplorable pour les victimes, qui sont en attente d'un cadre plus protecteur. L'introduction, au cours de la navette, de la « clause de Roméo et Juliette », doit permettre d'éviter une telle censure. Il s'agit de prendre en compte dans notre droit ce qui peut être qualifié d'« amours adolescentes » caractérisées par un faible écart d'âge entre une personne mineure et une personne majeure. Avec l'adoption de ce texte, les choses seront donc claires : toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans sera considérée comme un viol. Dans le cadre d'une relation intrafamiliale, tout acte sexuel commis sur un mineur par un proche ayant une autorité de droit ou de fait sera désormais qualifié de viol incestueux. Le débat parlementaire n'a pas seulement permis de modifier des curseurs d'âge, si importants soient-ils. Sur notre initiative, complétée par le travail de l'Assemblée nationale, il a également permis de préciser notre droit, ainsi rendu plus proche de la réalité que vivent encore de trop nombreuses victimes. C'est ainsi que nous avons introduit, dès la première lecture au Sénat, la prescription glissante pour les cas de crimes sériels. L'Assemblée nationale s'en est emparée, et je me réjouis que la disposition ait été conservée. C'est également le Sénat qui a proposé l'introduction des rapports bucco-génitaux dans la définition légale du viol, réparant un oubli dommageable dans notre droit. l'initiative de notre rapporteur Marie Mercier, la commission des lois a amélioré le texte en modifiant par exemple la nouvelle infraction pénale introduite à l'Assemblée nationale visant à réprimer le fait, pour un majeur, de demander à un mineur l'envoi d'images pornographiques de lui-même. Notre commission des lois a fait le choix d'élargir la protection des mineurs en prévoyant que cette nouvelle infraction concerne l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de 15 ans. De la même manière, nous avons fait le choix, en commission, d'élargir la protection garantie aux mineurs dans les cas de « sextorsion ». Ce délit, qui consiste, pour un majeur, à extorquer la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique d'un mineur, permettra de protéger l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de 15 ans. La peine sera quant à elle aggravée si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou en bande organisée. Mes chers collègues, le texte tel qu'il nous revient en deuxième lecture est- je le crois -un texte d'équilibre, adapté aux enjeux de notre temps. Ce sujet difficile peut demain concerner chacun de nos enfants. Ne nous faisons pas d'illusions : la réponse pénale que nous organisons aujourd'hui est certes un élément essentiel de la lutte contre les crimes sexuels commis sur les mineurs, mais elle n'en constitue qu'une partie. Le reste du travail, complexe, doit mobiliser l'ensemble de la société, dans les milieux associatifs, auprès des familles, dans les écoles, les collèges et les lycées, sans oublier internet, qui constitue sans aucun doute le grand enjeu de demain. À la place qui est la nôtre dans cet hémicycle, nous avons fait notre devoir ; je crois que nous pouvons collectivement en être fiers. L'unanimité qui a prévalu en première lecture, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, nous oblige. Le travail se poursuit cet après-midi. Nous le devons à toutes les victimes,

jeunes victimes : la vie d'un nombre important de personnes- des centaines de milliers, peut-être même davantage, dans notre seul pays -, a été abîmée, gâchée ou ruinée par des personnes qui se devaient au contraire de protéger et de faire grandir. Rappelons que, selon un sondage, près de la moitié des victimes de viol dans l'enfance auraient fait par la suite une tentative de suicide. Nous ne le dirons jamais assez : les viols sont une honte pour notre pays et, plus largement, pour toutes les nations de ce monde qui les acceptent sans les punir. En France, environ deux enfants par classe sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité ; 81 % des violences sexuelles commencent avant 18 ans, la première agression survenant en moyenne à 9 ans, au moment du CM1 Dans 94 % des cas, elles sont commises par des proches. Depuis des années, une prise de conscience collective s'est opérée grâce aux professionnels de la prévention, de la santé et de la répression, grâce, aussi, à une évolution des mentalités- il n'est plus interdit de tout interdire, au contraire : il est même parfois recommandé d'interdire ce qui doit l'être.

La parole des victimes s'est libérée et rien ne doit arrêter ce mouvement. Selon le juge Édouard Durand, le passage à l'acte de l'adulte est une perversion du besoin affectif de l'enfant. En aucun cas un enfant ne peut être consentant à une relation sexuelle, et il est bien que ce texte le dise.

J'ai aussi la conviction, depuis plusieurs années, que la lutte contre les violences physiques et sexuelles dépasse nos ego et nos clivages. Je suis fière que cette proposition de loi puisse constituer, en la matière, un remarquable pas en avant, et je pense que nous pouvons être collectivement fiers d'y avoir contribué, sur toutes les travées de cette assemblée.

femmes ! Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, grâce à nos débats, le texte a évolué et s'est profondément enrichi. Pour autant, à titre personnel, je reste réservée sur l'infraction autonome. Je crois toujours que nous devons insister sur l'absence de contrainte et non sur l'absence de consentement, car seul l'auteur est responsable de tels actes ; jamais un enfant ne peut consentir. Une seconde voie était constitutionnelle, consistant à respecter tant le principe de la présomption d'innocence que le principe d'égalité devant la loi. Je m'interroge aussi sur l'institution d'un écart d'âge de cinq ans permettant de ne pas criminaliser les amours adolescentes. les amours adolescentes. Cette clause telle qu'elle est aujourd'hui proposée crée en effet une entorse au principe que nous tentons de défendre. Malgré ces réserves, je suis convaincue que le texte que nous devons voter va dans le bon sens. Il répond aux préoccupations exprimées tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Nos travaux ont permis de dégager un consensus sur un certain nombre de principes je me réjouis par exemple de l'adoption de l'amendement visant à élargir la liste des infractions entraînant une inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes,

celles qui ont été votées à l'Assemblée nationale, l'instauration d'un seuil d'âge de 15 ans notamment- je l'ai moi-même toujours défendu. Il était important que la justice se focalise sur l'agresseur et non plus sur le comportement de la victime. Il est possible que l'agresseur ait utilisé la violence, la menace ou la surprise,

Albert Einstein disait : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » En l'espèce, nous avons tous, collectivement, essayé d'agir.

entre l'âge de la victime et l'âge de l'auteur. Vous parlez d'« amours adolescentes » ; mais savez-vous que l'âge moyen de la première relation sexuelle est de 17 ans et 6 mois pour les filles et de 17 ans pour les garçons ?

les personnes handicapées, mineures et majeures, dans nos débats, comme cela a été le cas lors de nos précédentes discussions. Je voudrais simplement rappeler la réalité de ce fléau à travers deux illustrations. Une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques de juillet 2020 démontre que la probabilité de subir des violences sexuelles est multipliée par deux pour les personnes handicapées.

ne peut améliorer le dispositif, nous en appelons à la mobilisation du Gouvernement pour enclencher une dynamique réelle sur les mesures de prévention la lutte contre ce fléau qui touche les personnes handicapées. Nous avançons aujourd'hui pour tous les mineurs ; c'est heureux. Le fléau réel cible particulièrement les personnes handicapées ; merci, monsieur le garde des sceaux, de redire

exclut de la liste des auteurs les frères et soeurs qui n'ont pas une autorité de droit ou de fait sur la victime, et qui peuvent être mineurs au moment des faits. Cet amendement vise à corriger cette erreur rédactionnelle en instituant que les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l'article 222-22-3 du code pénal, sans condition d'autorité de droit ou de fait.

la proposition de loi amoindrit son ambition et diminue la protection des mineurs victimes d'inceste. En effet, une autorité de droit ou de fait devra être démontrée, démontrée, alors même que les auteurs des faits criminels sont des membres de la famille de la victime. Cette faille favorisera l'impunité des agresseurs. Or il est essentiel d'éviter toute confusion et de rappeler que l'inceste est un interdit anthropologique.

sexuelle incestueuse. La rédaction actuelle- « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait

parfaitement neutre : il renvoie simplement au fait d'accomplir un acte, sans connotation de culpabilité. En l'occurrence, le texte ne prévoit pas que le mineur commet un viol. Il tend seulement à indiquer ce qui est factuellement exact, c'est-à-dire pénètre le corps de l'agresseur si celui-ci lui impose une fellation : cela ne fait évidemment pas du mineur un violeur, car il faut un élément moral

pénal n'auront pas forcément connaissance de nos débats et se demanderont quelle nuance le législateur a voulu introduire en distinguant l'acte de pénétration « commis » par le majeur de celui qui est « exercé » par le mineur. Ces considérations nous ont donc conduits à émettre un avis défavorable

Cet élargissement poserait un problème constitutionnel puisqu'il aboutirait à criminaliser automatiquement un rapport consenti entre, par exemple, un neveu et sa tante, même s'ils sont tous les deux majeurs. Par ailleurs, il pose problème au regard du principe de liberté sexuelle qui découle du principe de liberté individuelle.

? Prenez l'exemple d'un frère et d'une soeur qui auraient des rapports sexuels : si l'on ne s'interroge pas sur le consentement des deux partenaires, si l'on ne recherche pas l'existence d'un rapport d'autorité dont l'un des deux aurait abusé, qui devrait figurer dans le box des accusés ? Les deux partenaires devraient-ils être poursuivis devant les assises ? Au-delà des problèmes de principe qu'il soulève, le dispositif proposé paraît donc tout simplement non opérationnel.

incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse. Comme je l'ai expliqué par anticipation dans mon discours lors de la discussion générale, je comprends la volonté de certains de nos collègues d'être dans le mieux-disant pour la protection des mineurs, mais notre responsabilité est d'adopter des dispositions législatives qui soient applicables applicables en toutes circonstances et qui permettent de désigner sans ambiguïté le coupable et la victime. Si cet amendement était adopté, en cas de relations sexuelles incestueuses le

peut permettre à la justice de prendre une bonne décision. La commission n'est donc pas du tout favorable à cet amendement. Enfin, l'amendement n° 3, qui prévoit l'élargissement de la définition de l'agression sexuelle

D'ailleurs, pour compléter- si je puis me le permettre -les propos de Mme la rapporteure, l'article 222-23 du code pénal utilise le verbe commettre sans aucune confusion possible. On distingue bien le mineur, qui est la victime, de l'auteur. L'auteur commet un crime et, en l'occurrence, la victime peut commettre un fait. Je suis donc défavorable à votre amendement.

d'une enquête, on constate qui est l'auteur, qui est la victime, quelles sont les circonstances de l'espèce, etc. C'est seulement ensuite que l'on peut identifier si les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie sont réunis.

qu'il exerçait bien une relation d'autorité de droit ou de fait sur l'enfant. Depuis deux ans, nous essayons de rendre le droit simple simple pour les victimes, simple quant aux interdits qu'il pose dans la société et simple pour les praticiens du droit que sont les magistrats. Nous cherchons à éviter l'ajout de critères supplémentaires rendant plus difficile

proportionnalité. J'ai ajouté- madame la sénatrice, je tiens le document à votre disposition : « Ce n'est pas une question tranchée ; elle est délicate et mérite une vraie réflexion, un approfondissement de nos travaux. » J'ai travaillé, je suis revenu devant vous et je dis ce que j'ai à dire sur cette question.

Nous avons eu l'occasion de l'évoquer, le critère de l'écart d'âge, qui conduit à ce que la loi que nous sommes en train d'élaborer et de voter ne s'applique pas lorsque le mineur a 14 ans et le majeur 19 ans, ne nous paraît pas poser un interdit clair sur les relations sexuelles entre majeurs et mineurs.

et se rallier en fin de compte aux propositions que nous faisons, parce qu'elles sont les plus protectrices. En instaurant un écart d'âge, vous en revenez purement et simplement au seuil de 13 ans

la loi, l'interdit, et la matière légistique donnée aux juges pour agir. Enfin, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous dire que

Cependant, il est difficile pour un parquet de classer sans suite des faits, s'ils sont constitués, que le législateur aurait décidé de qualifier de crimes. Nous devons donc être cohérents avec nous-mêmes : nous ne pouvons pas qualifier certains comportements de crime, qui est l'infraction la plus grave, puis expliquer dans la minute suivante que certains des comportements visés ne posent en réalité pas de problème et ne doivent pas être poursuivis. Il nous appartient de définir des règles qui soient générales et impersonnelles et qui pourront s'appliquer à toutes les situations visées. Sur un plan que je qualifierais de plus politique, je signale également que le seuil de 15 ans assorti de l'écart d'âge de cinq permet en réalité d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé au Sénat en adoptant un seuil de 13 ans, puisque nous avions augmenté la protection des 13-15 ans. Nous devons être cohérents avec la position que nous avons adoptée, une position réaliste qui tient compte de l'existence de relations consenties entre des mineurs d'un peu moins de 15 ans et de tout jeunes majeurs. Parce que c'est la réalité de la vie

réglant ces questions une fois pour toutes ? Vous n'avez pas pris l'ombre de l'once d'un texte en la matière ! Je me permets de vous le rappeler, parce que la critique est facile, mais l'art est beaucoup plus difficile ... Pour le reste, la vie s'impose à nous.

sont établis ? Quand on veut être l'arbitre des élégances comme vous, on laisse au moins les interlocuteurs s'exprimer jusqu'au bout. Vous m'avez donné des leçons- vous adorez faire cela ! -depuis que nous nous connaissons d'ailleurs, mais il faut vous calmer,

Je le redis, je ne veux pas être le garde des sceaux qui renvoie aux assises un gamin de 18 ans et quelques jours parce qu'il a eu une relation avec une jeune fille. Pourquoi un écart d'âge ? Nous avions évoqué la notion de

effet, il existe en droit français le principe de l'opportunité des poursuites, en vertu duquel le parquet apprécie les circonstances de l'espèce avant de décider de renvoyer ou non tel ou tel devant la cour d'assises.

Je ne pense pas que vos propos, que je pourrais qualifier- je ne le pense pas vraiment -d'injurieux, soient très utiles pour éclairer notre réflexion.

contre les violences sexuelles commises sur les enfants. Avant cela, j'ai lutté contre les violences sexuelles commises sur les femmes, contre les agressions sexuelles, contre le harcèlement sexuel, contre la misogynie, contre le sexisme. Or, chaque fois

la liberté sexuelle ! C'est tellement mieux d'être empathique à l'égard de ces « amours adolescentes » entre quelqu'un de 14 ans et demi et quelqu'un de 19 ans ! Mais, toujours au nom

Puisque nous sommes en train de déterminer de nouvelles règles en matière de seuils d'âge et de circonstances pendant lesquelles une protection spécifique doit être accordée, il nous semble très important que

de continuer de travailler sur la vulnérabilité des jeunes qui se trouvent en situation de handicap. Néanmoins, je voulais lancer

un jeune majeur qui aurait une des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans, enceinte, par exemple, serait automatiquement l'auteur d'un viol. La loi n'imposerait pas de s'interroger sur le consentement de la jeune fille, ni même de se demander si le jeune majeur a abusé d'une quelconque autorité.

la loi pénale consacre déjà une circonstance aggravante dans certaines hypothèses de vulnérabilité, notamment en cas de handicap. Parfois, Parfois, dans certaines hypothèses, la loi facilite la preuve de la contrainte quand il y a une vulnérabilité inhérente à un handicap.

de ces violences faites aux femmes en situation de handicap. Nous avions alors mené de nombreuses auditions et nous avions adopté, à l'unanimité, une proposition de résolution

entre le majeur et le mineur, lorsqu'il s'agit de relations sexuelles obtenues en échange d'une rémunération, c'est-à-dire de prostitution, pour faire simple.

qui mobilise le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, mais également tous les directeurs d'établissement à caractère social, les commissariats et les gendarmeries ainsi que les juges pour enfants.

les auteurs de relations sexuelles sur des mineurs de 15 ans. Cela me paraît cohérent avec notre volonté commune de lutter contre la prostitution des mineurs.

nous reparlerons. Vous noterez néanmoins que ce texte vise à protéger les mineurs de 15 ans en fixant des règles de droit dérogatoires qui tiennent compte de leur vulnérabilité et de leur manque de discernement. L'adoption de votre amendement aboutirait à traiter tous les mineurs de la même manière, sans distinguer la situation du jeune de 17 ans et demi de celui de 12 ans. C'est très contestable. Je note également que l'achat d'actes sexuels auprès de mineurs est déjà réprimé par l'alinéa 2 de l'article 225-12-1 du code pénal, issu de la loi du 13 avril 2016 que vous connaissez bien, madame la sénatrice, visant à renforcer la lutte

puisqu'il créerait une double incrimination pour les mêmes faits. Il est bien sûr permis de s'interroger sur les raisons qui nous conduiraient à passer de trois ans d'emprisonnement- c'est la peine adoptée par la majorité socialiste en 2016 -à vingt ans de réclusion criminelle. Il convient donc de conserver une proportionnalité dans les peines que nous prévoyons et je doute que celle-ci serait assurée avec l'adoption de cet amendement. En outre, on note que la peine encourue est une contravention de cinquième classe punie de 1 500 euros en cas de recours à la prostitution d'un majeur. On passerait donc d'une peine de vingt ans de prison avec un mineur de 18 ans moins un jour, à une simple contravention dans le cas d'un majeur de 18 ans et un jour. Il n'est pas certain qu'un tel écart soit véritablement proportionné. Je retiendrai vraiment de votre amendement que nous devons lutter contre la prostitution en règle générale.

L'homme qui paie une jeune femme de 18 ans et un jour pour avoir des relations sexuelles s'expose à 1 500 euros d'amende. Le même qui a une relation sexuelle avec une jeune femme de 18 ans moins un jour, s'il la paye, encourt vingt ans d'emprisonnement.

pas rien ! En matière pénale, c'est toujours la même chose : certains pensent que pour complaire aux victimes, il faut prévoir des seuils qui ne sont jamais satisfaits. C'est, au fond, la surenchère dont je parlais tout à l'heure en disant

qu'un mineur de 18 ans qui se prostitue est considéré comme relevant de l'enfance en danger et de la protection de l'enfance. Un mineur de 17 ans et 9 mois qui se prostitue est un enfant en danger.

ce n'est en aucun cas celui que nous devrions avoir s'agissant de la protection globale des enfants de moins de 18 ans exposés aux clients de la prostitution. Je suis effectivement favorable à la pénalisation de tous

En revanche, on peut être d'accord sur le fait que protéger les mineurs de la prostitution et des clients est une exigence collective fondamentale.

en son nom et partage ses arguments. La souffrance des victimes ne s'efface pas. Pis, elle se révèle parfois tardivement, du fait de l'amnésie traumatique. Le régime de la prescription, s'il a évolué ces dernières années, continuera d'exclure de trop nombreuses victimes. Nous convenons, dans nos débats, du caractère souvent inintelligible du cadre législatif que nous posons. Si nous, législateurs, éprouvons la plus grande difficulté à énoncer la règle, comment nos concitoyens pourront-ils s'y retrouver ? Un cadre clair passe par l'énonciation d'interdits clairs : un adulte n'a pas de relation sexuelle avec un enfant et on ne doit même pas se demander si l'enfant a pu y consentir. Ce serait nier son essence même d'enfant et tourner le dos à notre impératif de le protéger. De la même façon, nous énonçons clairement les conséquences pour ceux qui feignent de reconnaître l'interdit : « La force de la justice vous poursuivra toute votre vie si vous commettez ces actes. Cette imprescriptibilité nous semble plus claire pour toute la société, plus juste pour les victimes et plus facilement opérante du point de vue technique. En outre, elle est psychologiquement plus acceptable que la prescription glissante qui consiste à devoir espérer, pour une victime, que son agresseur ait de nouveau commis l'irréparable avec une autre victime plus récente pour entrevoir une action en justice. Clarifions donc la situation en rendant imprescriptibles les crimes sexuels sur mineurs.

son encontre. Par définition, l'inceste se passe dans le huis clos des familles, il faut donc se préoccuper de la protection de l'enfant qui a déjà du mal à révéler

pour que soit statué très rapidement, en l'occurrence sous huitaine, sur la suspension des droits de visite et d'hébergement du mineur concerné.

d'envisager le fait que l'enfant ne soit plus contraint de résider avec l'auteur potentiel de l'inceste commis à son encontre.

les outils. Le droit de visite et d'hébergement peut déjà être tout à fait suspendu ou retiré en cas de motif grave tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment, et c'est heureux, en cas de mise en danger de celui-ci. Le procureur peut en effet saisir le JAF, mais ce n'est pas une obligation. Par ailleurs, concernant la non-présentation d'enfant, dans le cadre de l'opportunité des poursuites,

Je note, pour terminer, que l'amendement présente un défaut de cohérence. Dès le début de l'enquête préliminaire, le JAF serait saisi et pourrait fort bien décider de préserver les droits du parent mis en cause s'il estime que les accusations portées contre lui sont vraiment trop ténues et peu étayées. Or l'autre parent pourrait, malgré tout, décider de ne pas présenter l'enfant sans encourir la moindre poursuite, et ce pendant toute la durée de l'enquête préliminaire. On se demande donc à quoi servirait la saisine du juge si l'autre parent peut de toute façon décider de ne pas présenter l'enfant. On voit bien les abus qui pourraient se produire dans l'hypothèse d'un climat familial conflictuel, ce qui est malheureusement souvent le cas. Cela étant, à la suite de la lecture de cet amendement, j'ai bien conscience que nous sommes là pour sauvegarder

les enfants. À cet égard, je crois que ce texte, s'il est appliqué correctement, va faire avancer la cause

Le scrutin est clos.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

séance est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (texte de la commission n° 473,

la commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat le mardi 23 mars dernier est parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi, déposée par M. le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. L'accord ne fut, il est vrai, pas difficile à obtenir, tant les positions de nos deux assemblées étaient proches, l'Assemblée nationale ayant préservé les grands équilibres du texte et maintenu les apports du Sénat. La proposition de loi, je le rappelle, vise à introduire dans notre code de procédure pénale une nouvelle voie de recours garantissant à chaque détenu la possibilité de faire constater des conditions indignes de détention, afin qu'il y soit mis fin. Le détenu aura la possibilité de déposer une requête, examinée soit par le juge des libertés et de la détention, si la personne est placée en détention provisoire, soit par le juge de l'application des peines, s'il s'agit d'un condamné. Il appartiendra au juge de se prononcer sur la recevabilité de la requête, puis, s'il estime la requête fondée, de prendre une décision pour mettre fin aux conditions indignes de détention, après avoir accordé un délai à l'administration pénitentiaire pour y remédier par ses propres moyens. Le texte ouvre une nouvelle voie de recours sans créer un droit automatique à la remise en liberté, ce à quoi nous étions attentifs. Différentes mesures pourront être étudiées par l'administration puis par le magistrat, y compris le transfèrement dans un établissement moins occupé, sans que cette mesure ait vocation à être systématique. Sur mon initiative, le Sénat a notamment veillé à ce que le juge d'instruction, qui peut avoir connaissance d'éléments importants pour la prise de décision, soit mieux associé à la procédure. Le juge des libertés et de la détention devra ainsi le tenir informé s'il estime qu'une requête est recevable et pourra le consulter avant de prendre sa décision. À son tour, l'Assemblée nationale a apporté d'intéressants compléments au texte, sur l'initiative de la rapporteure de sa commission des lois, Caroline Abadie. Je note en particulier la disposition selon laquelle seraient déclarées irrecevables des requêtes successives présentées par un même détenu en l'absence d'élément nouveau. Cette précision devrait contribuer à éviter un usage abusif de la procédure, lequel aurait pu dégrader les conditions d'activité des juges des libertés et de la détention et des juges de l'application des peines, ainsi que nous en avions exprimé Il est également opportun d'avoir enserré l'appel dans des délais, cette mesure étant cohérente avec la manière dont ont été conçues les autres étapes de la procédure. Lorsqu'un détenu souffre de conditions indignes de détention, il convient qu'une décision soit prise rapidement, en première instance comme en appel. Je sais que certains ont pu regretter que la proposition de loi ait été examinée selon un calendrier très resserré. Sur un texte qui touche aux droits fondamentaux, il convenait cependant d'avancer rapidement. Au reste, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel nous avait donné jusqu'au 1 mars pour introduire dans notre législation ce nouveau droit de recours effectif. Cette date butoir ne pourra être tenue, mais l'initiative de François-Noël Buffet nous aura au moins permis de répondre à cette exigence constitutionnelle dans un délai aussi rapproché que possible. C'est vrai ! Je suis persuadé que l'entrée en vigueur du texte constituera une étape importante pour la garantie des droits fondamentaux dans notre pays, mais je suis également conscient qu'il ne suffira pas, à lui seul, à résoudre les problèmes constatés dans nos prisons. La promulgation de la loi ne nous dispensera donc pas de continuer à investir pendant encore de longues années dans la remise à niveau de notre parc pénitentiaire et de poursuivre l'embauche de personnels pénitentiaires afin d'améliorer durablement les conditions de détention. La parole est à M.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, instaurer un recours effectif tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, c'est une exigence constitutionnelle, mais c'est avant tout une question d'humanité. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir d'être rapidement parvenus à un consensus sur cette proposition de loi pour répondre dans les meilleurs délais au Conseil constitutionnel. À ce titre, je tiens à saluer l'initiative qui fut la vôtre, monsieur le président de la commission sur la base d'un travail que nous vous avions proposé en décembre dernier pour faire aboutir au plus vite cette modification législative devenue indispensable. doit évidemment protéger nos concitoyens et la société dans son ensemble, mais elle doit également, comme le rappelle à titre liminaire la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et à la prévention de la récidive. Or les peines exécutées en maison d'arrêt dans des cellules où s'entassent parfois plusieurs détenus, lesquels dorment sur des matelas à même le sol, sont totalement contre-productives. Plus elle désocialise et déshumanise, plus l'incarcération est un vecteur de récidive. Permettre aux personnes écrouées de contester leurs conditions de détention devant le juge judiciaire constitue une avancée significative, car la peine, en particulier la peine d'emprisonnement, doit avoir un sens. La prison ne peut pas être une privation de dignité. En cela, le recours effectif que nous avons conçu, dans une coconstruction efficace, que je tiens à souligner, constitue un dispositif cohérent, qui s'inscrira parfaitement dans notre droit. Cette proposition de loi nous permet de réformer notre droit dans le délai très contraint fixé par le Conseil constitutionnel. Aussi, je tiens à remercier la commission des lois du Sénat, tout particulièrement son président François-Noël Buffet, de son initiative. Je remercie également le rapporteur, Christophe-André Frassa, de son implication. Il me faut par ailleurs saluer le travail mené par la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale et par sa rapporteure sur ce texte, Caroline Abadie. Je ne peux que me féliciter de la qualité des échanges parlementaires sur cette question aux enjeux essentiels et des propositions constructives des deux assemblées, qui nous ont permis d'améliorer significativement le dispositif de ce recours effectif. Plus précisément, ce texte crée un nouvel article 803-8 dans le code de procédure pénale, qui pose le principe d'un recours effectif devant le juge judiciaire, et rappelle son existence dans un nouvel alinéa de l'article 144-1 du même code s'agissant des prévenus, ainsi qu'à l'article 707 pour les condamnés. Le magistrat compétent pour statuer sur les requêtes des personnes en détention provisoire sera le juge des libertés et de la détention. Pour les condamnés en exécution de peine, c'est au juge de l'application des peines qu'il reviendra de prendre une décision. Après avoir statué sur la recevabilité de la requête, le magistrat saisi pourra faire vérifier les allégations circonstanciées du détenu et, s'il estime la demande justifiée, il fixera le délai dans lequel l'administration pénitentiaire pourra mettre fin aux conditions indignes de détention, le cas échéant en transférant la personne dans un autre établissement pénitentiaire. Si les conditions indignes perdurent au-delà de ce délai, le juge pourra ordonner lui-même un transfèrement ou, pour les prévenus, la libération de la personne, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique. Pour les condamnés, il pourra prononcer une libération sous aménagement de peine si la personne est éligible à une telle mesure. Les travaux menés en coconstruction par les deux assemblées ont permis de rendre le texte initial plus lisible et notamment de préciser les délais de recours dont bénéficie la personne écrouée. Ce dispositif répond donc aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Il est à la fois clair, précis, efficace. Je suis parfaitement conscient qu'il ne peut être la seule réponse à l'amélioration des conditions de détention, objet de toute mon action depuis ma nomination à la tête du ministère de la justice. Il nous faut d'abord mener une politique plus volontariste de régulation carcérale, en poursuivant activement, en lien avec les chefs de cour et de juridiction et les services pénitentiaires, l'accompagnement de l'application des dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. en poursuivant la construction du programme immobilier pénitentiaire, dont j'annoncerai les derniers sites d'implantation dans quelques semaines, mon objectif est non pas d'incarcérer plus, mais de permettre des conditions de détention plus dignes. Pour cela, il nous faut renouveler le parc vieillissant et parfois vétuste et créer de nouvelles places de prison. Enfin, la dignité passe évidemment par le fait de donner aux personnes incarcérées la possibilité de se réinsérer, notamment par le travail. Je souhaite ainsi faire venir davantage d'entreprises en prison, et il m'est apparu essentiel d'instituer un véritable contrat de travail et des droits sociaux au bénéfice des détenus. Je reviendrai sous peu vous présenter ces nouvelles dispositions. La France ne doit plus être condamnée pour l'indignité de ses prisons. Cette proposition de loi ajoute un dispositif efficace dans l'amélioration des conditions de détention, dont nous pouvons collectivement nous féliciter.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous le savons, la France fait partie des États européens dont les prisons sont les plus encombrées et dont la population pénale augmente. En 2019, un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établissait que la densité moyenne des maisons d'arrêt en France était de 138 personnes pour 100 places opérationnelles, quarante-quatre de ces établissements ayant une densité supérieure à 150 %. Pour certains d'entre eux, le taux d'occupation pouvait aller jusqu'à 200 %, voire 213 %. Alors que le principe d'encellulement individuel est inscrit dans notre droit depuis la loi de juin 1875 sur le régime des prisons départementales, cette surpopulation chronique a de graves conséquences sur les droits et la dignité des détenus. Notre pays est d'ailleurs régulièrement condamné pour des conditions de détention contraires aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Prenant acte des divers arrêts et sanctions visant notre République, la proposition de loi présentée par notre collègue François-Noël Buffet a deux objets principaux le premier est de garantir à tous les détenus des conditions de détention compatibles avec le principe de dignité de la personne humaine ; le second est de créer une voie de recours effective lorsque la dignité du détenu est bafouée. Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l'ensemble des dispositions restant en discussion. Je souhaite néanmoins faire plusieurs remarques. En premier lieu, je regrette que, sur ce sujet, ce soit une proposition de loi qui vienne apporter une réponse aux injonctions qui sont adressées à la France et que le Gouvernement n'ait pas affiché de véritable ambition pour faire cesser une situation insupportable au pays des droits de l'homme. En second lieu, il est bien évident que l'adoption de cette proposition de loi ne résoudra pas, à elle seule, le problème posé par les conditions de détention dans notre pays. Elle ne nous dispensera pas non plus de poursuivre notre programme de construction et de rénovation de places de prison. Je veux rappeler que le Gouvernement s'est engagé à ouvrir 7 000 places d'ici à 2022 et à lancer des opérations pour l'ouverture de 8 000 places supplémentaires à l'horizon de 2027. Mon collègue Alain Marc, dans le cadre des travaux de la commission des lois, a régulièrement relevé le manque d'ambition de ce programme, qui se contente de prolonger des projets lancés par la précédente majorité, alors qu'il faudrait les amplifier. J'espère que vos annonces, monsieur le garde des sceaux, seront suivies d'effets concrets. concrets. Aussi, je souhaite insister sur la nécessité de ne voir ni retard ni mesures budgétaires affecter ou freiner la réalisation de ce programme immobilier. Avant de conclure, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance aux personnels pénitentiaires. une pensée toute particulière pour ceux de la maison centrale de Clairvaux, que vous avez rencontrés, monsieur le garde des sceaux. Ils remplissent une mission majeure, dans des conditions de travail souvent très difficiles. Mes chers collègues, reconnaître et respecter la dignité des détenus n'est pas une mesure de complaisance. Il s'agit d'une mesure indispensable pour faire de ces derniers des citoyens à part entière et leur permettre une vraie réinsertion dans le corps social. Cette proposition de loi représente une grande avancée pour notre démocratie. Le groupe Les Indépendants, particulièrement attentif au respect des droits fondamentaux des personnes, votera ce texte à l'unanimité. La parole

Les décisions rendues depuis des années sont édifiantes et font honte à notre pays. Comment encore accepter, au XXI siècle, qu'un juge doive imposer de vérifier que chaque cellule dispose d'un éclairage et d'une fenêtre en état de fonctionnement fonctionnement ou demander à l'administration pénitentiaire de trouver un autre moyen de servir les repas que de déposer les barquettes à même le sol ? Ce n'est pas nouveau. C'est, hélas ! une réalité bien ancrée dans notre pays, et nous ne cessons de critiquer le sort réservé aux détenus dans les prisons françaises. Les chiffres de la surpopulation sont aussi alarmants : en moins de vingt ans, les prisons françaises sont passées de 48 000 à 72 000 personnes détenues. Si ce chiffre a récemment connu une légère baisse liée à la crise sanitaire, moins qu'au 1 janvier 2021 ce sont plus de 20 000 personnes qui sont encore détenues dans des établissements, dont le taux d'occupation est supérieur à 120 %, allant même parfois jusqu'à 200 %. Cette surpopulation carcérale est une constante des dix dernières années. Cette situation, nous ne pouvons pas prétendre la découvrir aujourd'hui. Déjà en 2018, ma collègue Esther Benbassa interpellait le Gouvernement sur les violences et les mauvais traitements que subissaient certains détenus à la prison de Villefranche-sur-Saône. La garde des sceaux d'alors ne lui avait formulé, hélas ! qu'une réponse reflétant le déni ordinaire des pouvoirs publics face à ce sujet si important, mais très peu traité par les médias ou porté par la société civile. Elle n'est pas la seule à avoir tenté d'alerter ces dernières années. Pourtant, ces nombreux appels sont restés lettre morte jusqu'aux décisions de la CEDH du 30 janvier 2020 et surtout du Conseil constitutionnel du 2 octobre dernier.

mixte paritaire ne vient pas s'attaquer à ce problème : il répond à l'injonction de la deuxième décision, celle du Conseil Constitutionnel, qui a considéré qu'il incombait au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge pour des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine.

de loi et nous y associer. Monsieur le garde des sceaux, selon votre prédécesseure, l'objectif du Gouvernement était que, « d'ici à la fin du quinquennat, des conditions de détention plus dignes et conformes aux engagements européens soient mises en place ». Le temps presse. L'action de notre chambre pour apporter sa pierre à cette transformation nécessaire du système carcéral vous oblige. Cette proposition de loi est une première étape. À défaut de présenter une mesure construite, forte, pour une lutte systémique contre les conditions indignes, elle permet une plus grande effectivité pour les personnes détenues de voir leur situation individuelle s'améliorer. Nous attendons toutefois une amélioration urgente des conditions de vie dans les lieux de détention,

Ce n'est pas en construisant de nouvelles prisons, sitôt construites, sitôt remplies, que l'on réglera le problème de la surpopulation carcérale. Tout à fait ! La réforme des lieux de privation de liberté reste un chantier ample et complexe, qui ne se limite pas à la question du foncier. le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte, lequel, à défaut de s'attaquer au problème général de la surpopulation carcérale, permet aux individus enfermés de faire valoir leurs droits face à ce naufrage.

au Parquet européen, le président de la commission des lois du Sénat a déposé, en février 2021, une proposition de loi s'en inspirant. Un mois et demi plus tard, Sénat et Assemblée nationale parvenaient sans peine à un accord sur ce texte lors de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 23 mars dernier. La proposition de loi de notre collègue François-Noël Buffet organise donc ce recours au juge judiciaire pour tous les détenus- qu'ils se trouvent en détention provisoire ou qu'ils soient condamnés -demandant à ce qu'il soit mis fin aux conditions de détention qui seraient contraires à la dignité humaine. L'article 803-8 nouveau, inséré dans le code de procédure pénale, permettra ainsi au juge de demander à l'administration pénitentiaire de vérifier la situation d'un détenu ayant apporté un commencement de preuve avec des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles, et d'apporter ses observations. Si le magistrat juge cette requête fondée, il fera savoir à l'administration les conditions de détention qu'il estime indignes et lui demandera d'y mettre fin en moins d'un mois. Si l'administration ne s'exécute pas, le juge pourra alors ordonner une mise en liberté, s'il s'agit d'un prévenu, un aménagement de peine pour un condamné ou le transfèrement de la personne- cette dernière possibilité devra bien évidemment tenir compte de la vie privée et familiale du requérant. L'Assemblée nationale a respecté le dispositif présenté par le Sénat en précisant néanmoins les délais successifs applicables à chaque étape de la procédure, y compris en appel, en soumettant la présentation de requêtes successives par un même détenu à l'existence d'éléments nouveaux afin d'éviter l'engorgement des tribunaux et en obligeant l'administration pénitentiaire à informer le juge des mesures prises. Nous en sommes tous conscients, la création de cette voie de recours indispensable ne saurait, à elle seule, redresser la situation que connaissent les établissements pénitentiaires de métropole et d'outre-mer de notre pays depuis de très nombreuses années. C'est la politique de déflation carcérale, menée par le Gouvernement et matérialisée par l'augmentation des crédits consacrés à la rénovation du parc pénitentiaire et au recrutement de personnel, par la construction de nouvelles places de prison et par la multiplication, chaque fois que cela est possible, des alternatives à l'enfermement, qui pourra en venir à bout. Encourageant le Gouvernement à poursuivre et à amplifier son action en ce sens, le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Elle n'empêchera pas non plus l'entrée dans une délinquance profonde que peut provoquer un passage en détention. Elle ne permettra pas non plus de lutter contre l'insalubrité carcérale, qui touche près de trente-cinq établissements pénitentiaires français, selon l'Observatoire international des prisons. Pour cela, il faudra du temps et de la volonté politique. Nous y veillerons. À ce terrible constat, s'ajoutait celui de l'impossibilité, dans notre droit, de signaler ces conditions et donc de les faire cesser. C'est là tout l'intérêt de cette proposition de loi. Je remercie le président de la commission des lois de l'avoir déposée. En créant un droit de recours effectif pour les prisonniers, ce texte permet à la France d'être en conformité avec ses engagements internationaux. C'est à ce titre que nous soutiendrons les conclusions de cette commission mixte paritaire. paritaire. Pour être efficace, ce recours devra nécessairement être rapide, ce que ne garantit pas le texte. Nous serons donc particulièrement vigilants quant à son application. Enfin, la création de ce recours nous donne l'occasion de réfléchir plus largement à l'incarcération et à ses conséquences dans le parcours des délinquants. Pensons à d'autres types de peines, sans remettre en cause le principe de l'incarcération. Interrogeons-nous sur les causes de la délinquance et ses motifs, notamment quand un cinquième des détenus est incarcéré pour une infraction liée aux stupéfiants.

eux sont détenus dans un des six établissements pénitentiaires spécialisés, beaucoup se trouvent dans les quartiers pour mineurs des prisons, où il n'est pas rare qu'ils subissent les mêmes conditions matérielles indignes et vétustes. Et que dire de l'intervention éducative continue quand les mineurs peuvent attendre plus d'un mois avant de voir un premier professeur

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel a décidé, le 2 octobre dernier, que le Gouvernement devait produire une loi, avant le 1 mars 2021, permettant aux personnes placées en détention provisoire de faire respecter le droit à être incarcéré dans des conditions dignes. Nous sommes Nous sommes aujourd'hui le 25 mars, et le texte qui arrive en bout de course n'est pas d'initiative gouvernementale, mais sénatoriale. Le travail est donc fait, et vous conviendrez, monsieur le garde des sceaux, qu'il était plus que temps : cette injonction du Conseil constitutionnel fait suite à un certain nombre de condamnations de notre pays par les instances européennes pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Et nous oublions souvent que des conditions de détention indignes sont synonymes de conditions de travail extrêmement dégradées pour nos personnels pénitentiaires Vous avez coutume de rappeler, en référence à Albert Camus, qu'« une société se juge à l'état de ses prisons ». Tout à fait ! La proposition de loi que nous allons définitivement adopter aujourd'hui vient, comme une piqûre de rappel, nous signaler que l'état de nos prisons n'est pas reluisant. Ce n'est ni de votre

nous alertons régulièrement, notamment lors des dernières grandes réformes de la justice, sur les problèmes structurels des prisons françaises, dont celui de la surpopulation carcérale que nous ne parvenons pas à enrayer. Il s'agit de l'une des causes principales des conditions de détention non conformes à la dignité humaine. Cela met surtout en lumière une ambition carcérale réduite à la détention de détenus, au détriment d'une véritable réflexion sur le sens de la peine et d'une politique de réinsertion ayant les moyens de ses ambitions. Votre idée de suppression des réductions de peines automatiques pourrait commencer à avoir du sens si les détenus avaient effectivement accès aux activités éducatives de réinsertion, aux formations et à l'emploi. Il n'en est rien, ou si peu aujourd'hui, comme l'a souligné récemment la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot. Nous souscrivons à cette proposition de loi, mais notre vote s'accompagne d'une forme d'amertume devant le retard accumulé sur cette question. Malheureusement, nous avons la conviction que cela ne changera pas grand-chose au regard des obstacles dressés sur le parcours du détenu, avant même le dépôt d'un recours, lorsqu'il estimera indignes ses conditions de détention. Cela fait beaucoup.

le maintien des liens familiaux- quand la personne est prévenue -ou encore la sauvegarde des autres droits fondamentaux, tels que le droit à la santé si la personne est engagée dans un parcours de soin, ou encore le droit à la réinsertion pour les personnes qui suivent une formation, travaillent ou préparent un projet d'aménagement de peine cela fait dire à l'OIP que, « s'il représente une avancée par rapport à l'existant, le dispositif adopté reste très largement insatisfaisant ». Notre collègue, M. Sueur, a tenté en vain de vous soumettre des amendements visant à améliorer le dispositif de transfèrement, mais aucun n'a été adopté,

Quel sens donner à ce texte ? Il devrait, selon nous, être un point de départ à une réflexion d'envergure sur la décroissance carcérale à engager d'urgence, seule réponse qui vaille pour lutter efficacement contre les conditions de détention indignes

le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici réunis à nouveau autour de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention après son passage en commission mixte paritaire, chargée, le 23 mars dernier, de trouver un compromis.

Il s'agit bien évidemment du respect des droits fondamentaux, mais pas seulement. C'est également la sécurité, tant celle des détenus que celle des personnels, et les conditions de travail de ces derniers qui sont en jeu.

Prévoir une voie de recours, c'est très bien ; améliorer les conditions de détention pour qu'on n'en ait plus besoin, c'est mieux ! C'est vrai ! Mais je sais que cette mission est extrêmement complexe, monsieur le garde des sceaux, et que le piteux état de nos prisons ne date bien évidemment pas de votre prise de fonction. Pour remédier au problème structurel de surpopulation carcérale, la France se doit d'adopter une réforme d'ampleur visant à rénover nos établissements pénitentiaires et à enfin disposer d'un nombre de places équivalent à celui des hommes et des femmes détenus aujourd'hui en France. C'est la raison pour laquelle nous invitons le Gouvernement à maintenir ses engagements visant à ouvrir 7 000 places d'ici à 2022 ... Nous y arrivons ! ... et à lancer les opérations pour l'ouverture de 8 000 places supplémentaires à l'horizon de 2027. La mise en oeuvre de ces objectifs devrait contribuer à améliorer une situation qui fait honte à notre pays. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste soutiendra sans réserve le texte adopté par la commission mixte paritaire. La parole

sans prendre en compte, ni en première lecture ni lors de la commission mixte paritaire, ce qu'ont dit et écrit à la fois l'Observatoire international des prisons

que je ne comprends toujours pas pourquoi un certain nombre d'amendements que nous avions proposés n'ont pas été adoptés, à aucun stade de la procédure.

... Pour ce qui est des délais, rien ne change. Pour ce qui est des conditions dans lesquelles la requête pourra être

deuxièmement, la mise en liberté- s'il s'agit de détention provisoire - ; et, troisièmement, un aménagement de peine. Nous avions proposé un ordre différent : refus

le groupe Les Républicains se félicite de ce qu'un accord ait pu être trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Je tiens à saluer particulièrement François-Noël Buffet, président de la commission des lois et auteur de cette proposition de loi d'initiative purement sénatoriale et transpartisane, ainsi que le rapporteur, Christophe-André Frassa. Leur travail honore, une fois de plus, le Sénat. Les travaux de notre assemblée ont été sérieux, comme de coutume. Ce n'est donc pas une surprise si nos collègues de l'Assemblée nationale ont conservé les dispositions de fond de ce texte. La proposition de loi tire les conséquences d'une récente décision du Conseil constitutionnel. Cette dernière fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France pour conditions indignes de détention de détenus. Le Conseil constitutionnel avait alors déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale et demandé au législateur de garantir aux personnes placées en détention la possibilité de saisir le juge par rapport à des conditions de détention qui porteraient atteinte à leur dignité. L'inaction du Gouvernement en la matière, malgré l'échéance du 1 mars fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 octobre 2020, a conduit le Sénat à proposer un texte permettant de concilier à la fois le droit à des conditions dignes de détention et la nécessité de garantir la sécurité des Français. Grâce à cette initiative du Sénat, notre droit sera bientôt mis en conformité avec les normes internationales. La France évitera ainsi d'éventuelles condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, voeu qui vous semble cher, monsieur le garde des sceaux. Pour la première fois, les requérants disposeront d'une voie de recours effective pour faire cesser ces conditions de détention indignes, ce que ne permettent pas actuellement les seules procédures de référé. Grâce au travail du rapporteur sur le texte, le Sénat a veillé à associer, avec pertinence, le juge d'instruction à la procédure instituée par la proposition de loi. Ce n'est pas sans importance, puisque près de 30 % des personnes incarcérées en France ont la qualité de prévenu et sont donc placées en détention provisoire. Notre assemblée a aussi amélioré la proposition initiale en complétant les possibilités de recours. Je pense, par exemple, au fait de faire appel de la décision du juge s'agissant de la recevabilité ou non de la requête formulée par le détenu. Elle a également précisé que l'obligation de statuer en appel dans un délai de quinze jours porte uniquement sur l'hypothèse d'un appel émanant du ministère public. Enfin, le requérant aura la faculté de demander à être entendu par le juge alors que la version initiale de cette proposition de loi laissait au seul juge cette faculté. Il est important de noter que la proposition de loi, du fait de ses dispositions équilibrées, ne consacre pas un droit absolu à la remise en liberté. Le groupe Les Républicains salue ainsi les garanties visant à éviter la libération inconsidérée d'individus dangereux ou susceptibles de récidiver, ainsi que les marges de manoeuvre laissées à l'administration pénitentiaire. Cependant, malgré la création d'un recours effectif, le problème de la surpopulation carcérale reste entier. Les matelas au sol ne sont pas acceptables dans un pays moderne. Cette année encore, la densité carcérale s'établit à 105 % et s'élève même à 122 % dans les maisons d'arrêt. La construction de nouvelles places de prison, régulièrement appelée de ses voeux par le Sénat, constitue la meilleure des solutions pour répondre aux conditions indignes de détention. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains

aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

du jeudi 15 avril 2021 après-midi. En conséquence, la proposition de résolution invitant le Gouvernement à envisager la poursuite de la procédure de ratification du CETA sera examinée avant la proposition de loi visant à garantir effectivement le droit à l'eau par la mise en place